La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le programme de stabilité et l'orientation des finances publiques sur la demande de la commission des finances. La parole est d'abord à monsieur Gabriel Attal Ministre délégué chargé des Comptes publics. Monsieur le président. Monsieur le. Président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général madame la rapporteur général mesdames et messieurs les sénateurs. Avec ce programme de stabilité, nous vous présentons une trajectoire de redressement réaliste et déterminée de nos finances publiques. Le moment dans lequel nous sommes est un moment de bascule. Celui de la fin de l'ère de l'argent gratuit et de l'impératif désendettement de notre pays. Il y a 5 ans, le gouvernement présentait une amélioration très sensible de nos finances publiques, je le rappelle, grâce aux réformes enclenchées dès 2017 la France revenait sous les 3% de déficit et sortait de la procédure pour déficit excessif. Il y a 3 ans, la crise du Covid nous frappait de plein fouet. Et c'est dans l'urgence que nous avons dû agir pour que le pays ne s'effondre pas et l'économie notamment. Nous ne le regrettons pas un seul instant car c'était le bon choix oui. Notre dette a augmenté pendant la crise Covid. C'est une évidence mais oui c'était nécessaire, voire vital de protéger nos concitoyens et un certain nombre d'études montrent que si nous n'avions pas fait ce choix là la dette aurait augmenté dans des proportions encore plus importante. En plus des dégâts que nous aurions connu pour notre économie, des millions de Français qui travaillent, s'en est suivi, le plan de relance au soutien au sortir de la crise sanitaire pour relancer notre économie. Puis les mesures pour faire face à l'inflation et en particulier le bouclier tarifaire qui a permis d'économiser près de 200 euros par facture d'énergie. Tout au long de ces crises et de la réponse qui a été apportée par les gouvernements successifs, il n'y a eu qu'une seule ligne aux lignes de force. La protection des Français. Il y a eu une conséquence évidente, l'augmentation de la dépense publique. La dette a progressé de 16 points, passant de 97% du PIB en 2019 à 113% du PIB en 2021. Je tiens à préciser 2 choses. D'abord cette augmentation de la dette se situe dans la moyenne des autres États européens sur la même période que la nôtre. L'Allemagne a vu sa dette progressé de 10. L'Italie de 16. L'Espagne de 20 points le décrochage de la dette française par rapport aux autres pays de l'Union européenne a eu lieu bien avant cette période au moment de la crise de 2008. La 2ème chose. C'est que nous avons changé d'époque depuis avec. L'augmentation massive de nos taux d'intérêt. Ils étaient autour de 1% il y a moins d'un an, ils sont aujourd'hui de 3%. Face à cette envolée des taux face à ce renchérissement de notre dette. Je le dis clairement, nous sommes à un moment de bascule, celui de la fin de l'ère de l'argent gratuit celui où nous devons absolument reprendre le contrôle de notre dette. Reprendre le contrôle de notre dette pour rester indépendant. Reprendre le contrôle de notre dette pour garder le contrôle sur nos choix et nos choix sont clairs, soutenir la France qui travaille, mettre le paquet sur nos services publics et accélérer la transition verte de notre pays. À cet égard je veux revenir avec vous sur la publication de l'agence Fitch de vendredi dernier. C'est un sujet important sur lequel un certain nombre de questions ont été posées cet après-midi à l'occasion des séances de questions au gouvernement, notamment par le rapporteur général Husson, mais aussi par messieurs Ferrero et demi. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Fitch a en effet décidé de dégrader notre notation souveraine. Ah ah ah avec moins avec une perspective stable alors que celle-ci était crédité d'une note de double à sous perspective négative depuis près de 2 ans. Bruno Lemaire l'a dit, je veux l'affirmer à mon tour ne cédons ni au pessimisme, ni au fatalisme. Je, c'est notre capacité collective à maintenir la crédibilité financière de la France et je veux rappeler à cet égard que l'agence Moody's a fait le choix, la semaine précédente. De ne pas revoir la notation de la France qu'elle qu'elle a maintenus en double A, perspective stable. Les observateurs extérieurs croit toujours en notre résilience. Pourquoi. Parce que l'immense majorité des investisseurs et des analystes savent que les réformes structurelles que nous avons engagées vont continuer à produire leurs effets jusqu'à la fin du quinquennat. Je pense à la réforme de l'assurance chômage, je pense à la baisse des impôts de production, la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés et bien sûr à la réforme des retraites. Ces réformes concours à un objectif, construire une société du plein emploi, oui nous voulons bâtir une société du travail tout en prenant en compte les aspirations profondes de nos compatriotes qui souhaite travailler autrement, bénéficier de davantage de liberté dans l'organisation quotidienne et de davantage d'opportunités tout au long de leur vie professionnelle, c'est ce grand chantier que nous souhaitons ouvrir avec les partenaires sociaux pour construire ce nouveau pacte de la vie au travail. Annoncé par le président de la République. Si la crédibilité financière de notre pays reste forte, c'est aussi parce que notre détermination à rétablir les comptes publics et totale et pour ma part. Je vois d'abord dans la publication de l'agence Fitch la confirmation qu'il nous faut engager de manière encore plus résolu sur ce chemin et accélérer le désendettement de notre pays. Notre dette n'est pas gratuite, elle doit évidemment être remboursé en 2027 la charge de la dette, la charge d'intérêts de notre dette devrait s'alourdir de 10 milliards d'euros du seul fait de la remontée de moto. La conséquence de cette eau qui augmente de cette dette qui file c'est son poids qui s'alourdit bientôt le remboursement de notre dette sera à nouveau le 1er budget de l'État. Malgré ce constat sans appel, certains responsables politiques font croire qu'il existe un chemin qui consisterait à ne jamais rembourser. Mais je le dis clairement, la tentation de l'ardoise magique, c'est la certitude de la faillite. Arrêtons de nous tromper d'adversaire. Notre adversaire, c'est la dette pas le sérieux budgétaire la fin de l'argent gratuit ne fait que confirmer l'objectif qui est le nôtre, nous devons tenir nos comptes et nous le ferons avec plus d'ambition encore car notre situation nous le permet nous commencerons à rembourser notre dette, d'ici la fin du quinquennat et nous ramènerons le déficit des administrations publiques sous la barre des 3%. Je parlais d'accélération de notre trajectoire de désendettement, c'est ce qui compte c'est ce que contient le P. stable dont nous discutons aujourd'hui. Je vous rappelle dans le précédent programme de stabilité que nous présentions avec Bruno Lemaire l'année dernière. Nous prévoyons alors un déficit de 2,9% en 2027. Et un ratio de dette de 112 5 % en 2027 dans le programme de stabilité que nous vous présentons aujourd'hui, nous accélérons notre trajectoire puisque ce programme de stabilité prévoit désormais un déficit de 2 7 % en 2027 et un ratio de dette de 108,3% à à horizon 2027 c'est 4 points de moins que dans le précédent stable. Nous ne céderons pas au réflexe fiscal. Souvenons-nous des quinquennats précédents. Nous n'avons jamais fait ce choix car nous refusons le matraquage fiscal, nous refusons de faire payer la facture aux classes moyennes. D'abord je considère que l'on est au taquet, en matière d'impôts en France. Ensuite ce n'est pas aux Français de servir de variable d'ajustement aux soubresauts de l'économie mondiale depuis 2017, nous avons baissé les impôts des ménages de plus de 25 milliards d'euros et ce n'est pas maintenant au moment où l'inflation alimentaire grignote le pouvoir d'achat que nous allons augmenter les impôts. Le programme de stabilité que nous vous présentons prévoit donc une diminution du taux de prélèvements obligatoires. Ensuite nous poursuivons cette voie avec la ferme intention de réaliser des économies en 2024 et jusqu'en 2027. Dans certains secteurs, nous dépensons trop et j'ai d'autant moins de scrupules à le dire que je ne suis pas un ministre du Budget allergique à la dépense publique. Je l'ai déjà dit. La revue de dépenses que nous avons initiée avec Bruno Lemaire permettra d'entrer dans le détail de ces économies, mais nous savons d'ores et déjà que certains secteurs peuvent mieux faire. Nous avons d'ores et déjà engagés. Les efforts qui sont nécessaires. En ciblant davantage nos dispositifs je veux prendre pour exemple la ristourne carburant qui a coûté l'an dernier 8 milliards d'euros aux finances publiques qui a été remplacée par une une indemnité carburant ciblée sur les travailleurs modestes à 1 milliard d'euros. Nous sommes passés sur le carburant de 8 milliards d'euros à 1 milliard d'euros de la même manière. Bruno Le Maire a annoncé la sortie progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Merci. Dans le programme de stabilise. Qui vous est présenté. Le ratio de dépenses publiques sur PIB passera de 57,5% en 2022 à 53,5% en 2027, c'est 4 points de moins pour y parvenir, évidemment, des efforts seront nécessaires. Là aussi sont venus nous du précédent programme de stabilité que nous avons, que nous vous. Nous avons présenté avec Bruno Lemaire l'an dernier. Comment se décomposer alors les efforts. Nous prévoyons alors une baisse de la dépense en volume de l'État de 04% et de 0 5 % pour les collectivités locales. Dans ce programme de stabilité. Nous avons revu la charge de l'effort parce que nous avons écouté parce que nous avons entendu les parlementaires et notamment les sénateurs. Les associations d'élus locaux. La répartition de l'époque de l'effort a donc été modifiée dans ce programme de stabilité, nous passons d'un effort de. Moins 04% en volume pour l'État et moins 0 5 % en volume pour les collectivités locales un effort de moins 0 8 % pour l'État, avec un effort de moins 0 5 % pour les collectivités locales inchangé donc mais l'État fera donc dans ce programme de stabilité et je l'espère, traduit dans la prochaine loi de programmation des finances publiques davantage d'effort que les collectivités locales, ce qui n'était pas le cas dans la précédente trajectoire. Un secteur. Verra ses dépenses augmenter, y compris en volume, ce sont les administrations de Sécurité sociale, avec une augmentation de plus 0 5 % en volume ce qui. Satisfera je l'espère la rapporteure générale Doineau nous préservons l'hôpital public des économies qui sont nécessaires. Ce programme de stabilité n'est donc pas un programme d'austérité. D'abord, un pays qui consacrent plus de 50% de sa richesse à ces dépenses n'est pas un pays qui fait de l'austérité. Et ensuite, je le dis, nous n'avons jamais conduit une politique d'austérité depuis 2017 car c'est à la fois injuste et inefficace. a cédé à cette tentation. Cela s'est toujours soldée. De la même manière, plus d'impôts, plus de chômage, moins de croissance et plus de déficit à la fin. Nous assumons donc le sérieux budgétaire car être sérieux. C'est ce qui permet d'être ambitieux ambitieux pour nos services publics pour notre école notre police notre justice, notre armée pour lesquels nous avons engagé un réarmement budgétaire ambitieux pour notre hôpital public. Je le disais et nos soignants qui ont tant donné pendant la crise sanitaire et qui donne tant de leur temps. Aujourd'hui encore, je rappelle que cette année les moyens pour l'hôpital public dépasse les 100 milliards d'euros. C'est inédit dans l'histoire de notre pays. C'est l'engagement du président de la République et nous le tenons parce que notre pays en a besoin et parce que les Français l'attendent. où sont nos ambitions en matière de déficit. Je l'ai dit, mais nous n'abandons rien de notre ambition en matière d'investissements pour nos services publics. En 2027, je le disais, la dépense publique représentera encore 53,5% du PIB, un des, un pays qui dépense 53,5% de sa richesse à un impératif que chaque euro dépensé le soit au service des Français et au service de l'ambition de ce quinquennat refaire de nos services publics, les meilleurs services publics d'Europe Car la réalité. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est que parfois nos concitoyens ont l'impression de payer beaucoup d'impôts et le sentiment de ne pas toujours savoir à quoi ils Servent. Et moi je veux me battre pour ces Français qui ont l'impression de payer toujours plus. Et parfois d'avoir moi. Au fond je souhaite placer notre stratégie de réduction de notre déficit et de notre dette sous le signe de la confiance, confiance que les Français doivent retrouver dans l'impôt, confiance dans nos services publics qui sont notre priorité et que nous voulons hissé, je le disais au rang de meilleur service public en Europe, confiance dans le fait que chaque euro dépensé soit un euro utile mais aussi pour que chaque euro du soit un euros payés. C'est le sens du plan de lutte contre les fraudes que je présenterai dans les prochains jours. Maîtriser nos comptes pour ne pas renoncer à nos priorités, dire aux Français, à quoi sert leur argent, tout en leur demandant de nous aider de contribuer à l'employé mieux lutter sans relâche contre celles et ceux qui fraudent et qui sapent la confiance dans le pacte républicain. Voilà notre feuille de route voilà les combats à mener pour servir au mieux l'intérêt des Français et je suis convaincue que nous pourrons n'aura tous nous rassembler autour de ces combats, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à présent monsieur Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Lors du tout récent déplacement de notre bureau. De la commission des finances à Berlin et Francfort la semaine dernière. Nous avons le plaisir d'échanger très directement avec nos homologues allemands sur la réforme des règles européennes. De coordination budgétaire prévu par le pacte de stabilité et de croissance. le savez repose sur 2 principes essentiels, le 1er une meilleure prise en compte des investissements nécessaires pour répondre aux défis de demain. D'une part et 2ème principe une possibilité de différenciation des objectifs de réduction de la dette et du déficit en fonction de la de la situation réelle des pays. La réforme qui est en cours est à mes yeux éminemment nécessaire. Car nous devons en effet nous adapter les règles précédentes n'ont pas permis d'assurer une maîtrise durable des déficits et par ailleurs nos économies sont sortis beaucoup plus et, pour certaines très endetté à la suite des crises sanitaires puis énergétique et je crois que nous ne pouvons pas ignorer. Ni le réchauffement climatique, ni la. Nécessité de renforcer notre résilience, technologique, industriel et ou énergétique. L'approche retenue par les Européens d'appliquer les règles budgétaires en fonction des circonstances et me semble-t-il, une bonne approche. Mais elle implique que chacun respecte de grands principes majeurs. Tout d'abord que les trajectoires des finances publiques présentées soit construite sur des hypothèses crédibles et que les objectifs de maîtrise des comptes soit évidemment à la hauteur. Or, Monsieur le Ministre. Ne me semble pas être le cas du programme de stabilité que vous nous présentez. Il ne répond de mon point de vue à aucun des deux objectifs et fragilise donc. Notre parole. La part de la France par rapport à nos partenaires en 1er lieu je vais évoquer le scénario de croissance économique. S'agissant de la croissance du PIB en volume. Le gouvernement considère que le scénario qui l'avait présenté lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques reste inchangée. Comme cet Automne, ce scénario n'est malheureusement pas partagé par les gens conjoncturistes et paraît donc très optimiste. Ainsi, lorsque le gouvernement anticipe plus 1,7% de croissance par an en moyenne. Le consensus Forecast. Qui agrège des prévisions réalisées par une vingtaine d'institut. Anticipe pour sa part plus virgule 4% par an. Le principal écart c'est la consommation des ménages que le gouvernement veut voir évoluer de plus 1,6% par an et qui ne progressait selon les conjoncturistes que de 1,401,1 Ensuite vous avez Monsieur le Ministre, décidé de réévaluer très fortement votre estimation du déflecteur du PIB. Qui mesure l'évolution des prix des biens et services produits sur une année. Ce des flatteurs est un paramètre alors certes très technique mais absolument majeur de la trajectoire des finances publiques car il commande l'évolution du PIB en valeurs sur lequel est calculé le produit des impôts en clair. Plus des flatteurs est élevé, plus le PIB est élevé et plus les recettes publiques sont importantes. Sans d'ailleurs que le gouvernement ne documente les motifs de sa révision le déflecteur du PIB atteindrait ainsi 5,4% en 2023, se dit augmentation de près de points par rapport à ce qui était prévu, il y a quelques mois dans le projet de loi de programmation des finances publiques. En outre, là encore les conjoncturistes malheureusement pour le gouvernement, ne partage pas votre analyse, à l'instar du FMI et de la Banque de France qui retiennent eux le chiffre de 3%. Quelles sont les conséquences d'une telle révision, c'est finalement assez simple, il contribue à augmenter le PIB de 50 milliards d'euros en 2023, en comparaison. Du projet de loi de programmation, ce qui permet d'anticiper. Plus de 13 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Voilà qui constitue avouez-le une révision technique bien opportune pour qui voudrait présenter des ratios de dépenses publiques de déficit et d'endettement plus favorable la difficulté je viendrai c'est que l'ensemble de la stratégie d'amélioration des comptes publics que vous présentez repose sur une hypothèse qui n'est malheureusement ni documenté ni partagée par les conjoncturistes. Certes, la Commission européenne dans ses prévisions d'Automne envisager elle aussi hein des flatteur de l'ordre, 5% en 2023. Mais alors elle prévoyait dans le même temps une croissance du PIB bien plus faible et l'écart entre le PIB anticipé pour 2023 par le gouvernement et la Commission s'élève à plus de 30 milliards d'euros. En réalité, on a l'impression que le gouvernement a fait le choix pour la plupart des indicateurs économiques de retenir l'hypothèse la plus favorable, ce qui ne me paraît pas raisonnable. En ce qui concerne la croissance potentielle. Le gouvernement continue de l'évaluer à plus 1,35% par an. Une nouvelle fois un scénario qui n'est pas partagé par la plupart des conjoncturistes. Comme d'ailleurs le Haut conseil des finances publiques le déclare le scénario de croissance potentielle me paraît trop élevé d'autant plus qu'ils reposent sur l'hypothèse selon laquelle ne économie fonctionnerait actuellement en dessous de ses capacités. Pour tout dire les enquêtes et les difficultés à recruter actuellement ne conduise à en douter. En conséquence, Monsieur le Ministre ce scénario macroéconomique que vous présentez me paraît reposer sur un ensemble d'hypothèses trop favorable. Trop optimistes. Trop peu documentés et en définitive trop fragile. Cela n'est pas de nature à asseoir la confiance dans le cadre de notre dialogue avec la Commission européenne et nos partenaires. J'en viens maintenant au 2ème point la trajectoire des finances publiques que vous présentiez. Depuis quelques jours les ministres en disent tout le bien qu'il faudrait en penser elle montrerait un effort plus important de maîtrise des dépenses et des que la France s'apprête à réduire son déficit et sa dette dans des délais qui était jusqu'ici inespérée malheureusement là encore la pratique la réalité me paraît bien. Tout d'abord je l'ai dit tout à l'heure en renvoyant son scénario revoyant son scénario macroéconomique. Le gouvernement prévoit que le PIB en valeur soit supérieur en 2027 de excusez du peu, 70 milliards d'euros par rapport à ce qui était envisagé il y a quelques mois dans le projet de loi de programmation. Dans ce contexte, les recettes publiques augmenteraient mécaniquement d'un peu plus de 33 milliards d'euros sans aucune mesure nouvelle. En effet, le gouvernement annonce des baisses d'impôts pour les classes moyennes dans l'avenir. Monsieur le Ministre, vous l'avez fait, mais je n'en trouve aucune trace dans le programme de stabilité en conséquence la prévision de recettes. Paraît extrêmement fragile. Ce qui est plus sûr. Par contre, c'est la prévision d'évolution des dépenses qui montrent une augmentation d'environ 30 milliards d'euros en 2027 par rapport à la cible présenté là encore il y a quelques mois à la fin de l'année 2022 dans le. La loi de programmation des finances publiques sur cette hausse. Je veux faire deux alertes majeures. D'abord 12 milliards environ correspondent à l'augmentation de la charge des intérêts de la dette qui constituerait, vous le savez malheureusement le 1er poste du budget de l'État. Pour le reste entre 17 et 18 milliards d'euros. Ça correspond à une hausse des dépenses ordinaires, je le rappelle, c'est-à-dire hors mesures de crise. Ainsi, par rapport au projet programmation les dépenses ordinaires sont prévus pour augmenter et malheureusement tant en valeur qu'en volume. Alors que le projet de LPFP que nous avons mis à jour lors du vote de la loi de finances pour 2023 prévoyait une augmentation des dépenses ordinaires de 0 7 % par an en moyenne. Celle-ci s'établit désormais vous À quoi seront consacrés ces crédits supplémentaires sur les dépenses ordinaires. Le programme de stabilité ne le dis pas et on se demande d'ailleurs bien. Où se trouvent les 5% d'économies demandées par la Première ministre aux différents ministères. Enfin, j'observe que si la loi de programmation avait été adopté au mois de décembre. Les objectifs inscrits en dépenses serait déjà dépassé. Le temps passe vraiment vite. En outre, j'ai entendu notre ministre de les comédies. Et le ministre des Comptes publics. Dire qu'ils avaient entendu les collectivités locales, vous l'avez rappelé il y a quelques instants et que le programme de stabilité prévoyez désormais un effort plus important de la part de l'État, comparativement, celui des collectivités territoriales. j'ai un peu cherché mais. Rien ne permet de le constater dans le programme de stabilité qui ne comporte aucun développement aucun tableau aucune donnée permettant d'apprécier la trajectoire de dépenses des différentes catégories d'administration sur la période 23 27. Nous en sommes pour l'instant au niveau des paroles et de l'incantation. Je demeure, ça ne va pas vous surprendre cohérent avec la ligne que nous avions tenu lors de l'examen du projet de programmation en effet la trajectoire des dépenses qui étaient proposés n'était ni assez ambitieuse ni documenté note de par ailleurs que je ne suis pas le seul à douter de la capacité du gouvernement à mener les réformes. Structurelles nécessaires pour la France puisque la baisse toute récente de notation par l'agence Fitch en constitue, me semble-t-il au moins une preuve supplémentaire. J'en viens enfin à la question du déficit et de l'endettement public. J'observe en effet que le programme de stabilité prévoit une amélioration du déficit public d'environ 4 milliards d'euros en 2027 par rapport à la trajectoire inscrite au projet de loi de programmation, c'est-à-dire environ 0 2 % de plus de points de PIB et donc un déficit qui s'établirait désormais à 2 7 % du PIB plutôt que de. Toutefois, ces bons résultats comptables repose sur l'hypothèse d'une progression plus rapide des recettes que les dépenses et donc sur un scénario macroéconomique qui nous paraît tout à fait contestable. En conséquence si le scénario d'une augmentation des dépenses, a de sérieuses chances de se réaliser, celui d'une hausse des recettes dans l'ampleur prévues par le programme de stabilité reste très incertain. En conclusion, ce programme de stabilité repose sur un scénario macroéconomique qui nous paraît trop optimiste et fragile s'agissant des finances publiques, il présente à la fois une trajectoire de recettes fondé sur une révision du des flatteur qui ne fait pas consensus et une accélération des dépenses plus importantes que c'est le prévue au projet. Programmation des finances publiques. En définitive, l'amélioration du déficit et de l'endettement apparaît à la fois très très limitées et incertaine dans ces conditions, le programme de stabilité ne nous paraît pas à la hauteur de nos engagements européens et il a affaibli la France auprès de ses partenaires. Je vous remercie. ensuite au président Claude Raynal, président de la commission des finances. Le truc. C'est pas évident. Merci de vos applaudissements chaleureux. Chers collègues. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur général madame la rapporteur général. Mes chers collègues. La loi organique relative aux lois de finances impose au gouvernement de transmettre le programme de stabilité, le programme national de réformes au plus tard 15 jours avant leur présentation à la Commission européenne. Afin qu'il puisse donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je regrette que comme chaque année, le gouvernement ne respecte pas le calendrier fixé et que cette année nous ne disposions même pas du programme national de réformes et du rapport d'orientation des finances publiques qui aurait dit, nourrir nos échanges. Suscitant rappeler notre débat s'inscrit dans un contexte particulier puisque comme chacun le sait, la dernière loi de programmation des finances publiques n'a pas été adopté. Le nous a indiqué. Hier, que l'Assemblée nationale examinera à nouveau en juillet. Cet exercice est aussi renouveler puisqu'il rompt avec la période de la crise sanitaire caractérisé, d'une part. Par un très fort niveau d'incertitude en matière de prévisions macroéconomiques. Et d'autre part par la suspension des règles du pacte de stabilité de croissance. Désormais, même si la crise énergétique et les risques financiers restent. L'exercice de prévision macroéconomique devrait devenir un peu plus fiable et ensuite peut-être surtout des règles budgétaires européennes. Nous l'espérons. En tout cas, réformée vont de nouveau trouver à s'appliquer à compter de 2024. Le programme de stabilité pour les années 2023 à 2027 réitère la prévision de croissance du PIB en volume du projet de loi de programmation à l'époque et comme actuellement le Haut conseil des finances publiques, la Commission européenne et les conjoncturistes avaient jugé le scénario propos optimistes. J'observe que le Haut Conseil renouvelle son message de prudence, en particulier en ce qui concerne l'estimation de la croissance potentielle et indique notamment que l'augmentation de l'emploi. Total paraît surestimé d'ailleurs de son côté l'OFCE, estime que l'année 2023 malheureusement devrait être l'année du retournement du marché du travail. Lors de l'examen du projet de loi de programmation. Une bataille s'est engagée entre le gouvernement et la majorité sénatoriale concernant la trajectoire à suivre en dépenses. Je note que le gouvernement manque de transparence en ne permettant pas de distinguer ce qui est dans sa trajectoire relève de la fin des mesures de soutien temporaire et des dépenses courantes. Il est sans doute là un point traiter pour rendre plus lisible nos débats budgétaires. La trajectoire de dépenses du programme de stabilité corrigé de l'inflation reste dans les grandes lignes comparable à celle proposée lors du projet de loi de programmation. Elle implique donc de réaliser d'importantes économies par rapport à la croissance tendancielle. Qui ne sont pas davantage documenté aujourd'hui qu'hier. Vous attendez, je crois, enfin en tout cas on l'a lu à la presse que les ministères vous indique comment il pourrait réaliser à peu près 5% d'économie. On sait néanmoins déjà sur quoi. Le gouvernement a fait porter les efforts les dépenses sociales avec une volonté plus budgétaire qu'autre chose d'attaquer le système de retraite n'y revenons pas ici le système d'indemnisation du chômage et demain comme annoncé, les minima sociaux. Au dollar. On sent le gouvernement prêt à courir un peu tous les lièvres à la fois pour mettre en scène une recherche d'économies. Récemment vous avez lancé monsieur le ministre. Une initiative, vous l'avez d'ailleurs rappelé à l'instant pour savoir si l'on en avait pour son argent. Quand on paye ses impôts. Comme si au consentement à l'impôt à la citoyenneté à la participation à un modèle social patiemment construit pouvait se substituer pour chaque individu, la formule thatchérienne bien connu. I want my money Back. Magnifique pour un prof d'anglais. Vous avez fait savoir. Qu'un accouchement coûterait 2600 euros à la communauté nationale, mais combien rapporte à la nation une vie mise au monde par l'hôpital public. Nous le dire ferez-vous preuve du même exercice de transparence en ce qui concerne les aides publiques versées aux entreprises et d'ailleurs aussi le rapport au collectif. Le programme de stabilité reste sur ce point dans la droite ligne de la politique gouvernementale, il n'y aura pas de mesures nouvelles en prélèvement obligatoire d'ici 2027 ou plutôt il y en a, ce seront des baisses d'impôts, vous avez effectivement un effet et vous l'avez rappelé promis récemment de baisser les impôts des classes moyennes sans préciser là non plus. Quels étaient vos intentions. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'une telle annonce rassure nos partenaires. Non plus que nos prêteurs au final j'observe que ce programme de stabilité répond au schéma habituel. Un scénario macroéconomique optimiste et des objectifs de baisse des dépenses très élevées. Je ne partage pas, vous le savez ces orientations, mais à ce stade, je me rassure. Elles ne sont pas véritablement crédible. Merci. La parole est à présent à Madame. Élisabeth Doineau, rapporteur général de la commission des affaires sociales.

Madame la présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur, chers collègues. La commission des affaires sociales ne va pas être plus indulgente que la commission des finances, je le regrette monsieur le Ministre, mais il en est ainsi. En fait les hypothèses macro-économiques sont. Optimistes comme ça a été dit, je ne reviendrai pas longuement sur le regard que porte le Haut conseil des finances publiques. À propos de ces hypothèses. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire lors de différents. Comment. Regards sur les, les différentes lois précédentes, le Haut Conseil considère que la prévision de croissance effective est effectivement très élevé. Elle est de 1,7% en moyenne sur la période 2025 2027. notamment pour ce qui concerne la hausse prévue de la consommation. Le Haut conseil doute également des hypothèses retenues en matière de croissance potentielle qui suppose des gains de productivité sensiblement plus élevé que ce que laissent attendre les tendances récentes et une augmentation de l'emploi total qui paraît surestimé. Alors au-delà de l'avis du Haut Conseil. Monsieur le Ministre, comment ne pas retenir l'avertissement que constitue la récente dégradation de la note de la dette française de double à double à moins par l'une des principales agences mondiales de notation Fichte. Alors. J'ai eu l'occasion ce matin de voir la chronique de Bertille Bayart dans Le Figaro. Elle dit tout le monde se fiche de Fitch, apparemment c'est un peu votre idée puisque vous vanter la la notation de l'agence Moody's hein qui vous semblent plus correct par rapport à l'appréciation qui pourrait être porté sur les comptes publics. Mais. Vous pourriez d'ailleurs nous préciser. Monsieur le Ministre, si vous anticipez des conséquences de cette évolution pour les conditions de financement des administrations publiques. C'est en tout cas sur la base de ces incertitudes qu'il convient de lire les prévisions du gouvernement relative aux administrations de Sécurité sociale, ce qu'on appelle communément les assauts. Qui figure dans le programme de stabilité en terme de solde. Il est prévu que les assauts consolident leur contribution positive au sol public au cours des années à venir, après un retour, je vous le rappelle dans le Vert en 2022, plus 0,3 point de PIB le seul de consolidé des administrations de Sécurité sociale s'établirait à plus 0,7 point de PIB dès 2023 et oscillerait ensuite entre plus 0, 6 points de PIB en 2024 et 0,9 point de PIB en 2027. Il est important, il me semble, de rappeler qu'il s'agit d'un seul de toute administrations de Sécurité sociale plus large, donc que le périmètre des lois de financement de la Sécurité sociale, qui je vous le rappelle sont pas dans le même état. Ce solde positif et d'ailleurs largement tirée par des organismes en dehors de ce périmètre. La cadette en tout 1er lieu hein qui, qui est l'amortissement de la dette puisque l'amortissement de la dette sociale est enregistré comme un bénéfice, ce qui est assez paradoxal. L'assurance chômage sous l'effet de la diminution du nombre de demandeurs d'emploi dont l'ampleur devra tout de même être vérifié mais dont on se réjouit je pense les uns et les autres et les organismes complémentaires de retraite notamment l'Agirc-Arrco. À l'inverse, même après la réforme des retraites, les régimes obligatoires de base de sécurité sociale devraient, eux, rester en déficit sur l'ensemble de la période. Couverte par ce programme de stabilité ainsi l'annexe du récent collectif social prévoit une dégradation des comptes dans les années à venir avec un déficit consolidé qui passerait de 8,2 milliards d'euros en 2023. Un peu plus de 13 milliards d'euros en 2025 et 2026. Dans ces conditions, monsieur le Ministre, comment gérer cette nouvelle accumulation de déficit alors même que le plafond de transfert à la cadette a été atteint. Envisagez-vous de demander au Parlement de nouvelles autorisations de transfert à la cadette à court ou à moyen terme. S'agissant de l'évolution des dépenses publiques. Je relève que le gouvernement prévoit un fort dynamisme des dépenses de la Sécurité sociale. Et vous l'avez précisé, Monsieur le Ministre, malgré l'extinction progressive des dépenses exceptionnelles liées à la crise épidémique. Mais cette extinction devrait être plus con compensée par la progression des prestations sociales les liée à l'inflation, en particulier les pensions de retraite et les prestations familiales. Je conclurai en soulignant que les réformes structurelles, sur lesquelles s'appuie le gouvernement pour amorcer une trajectoire de désendettement concerne pour l'instant uniquement la sphère sociale qu'il s'agisse de la réforme de l'assurance chômage ou de la réforme des retraites et je souligne également Monsieur le Ministre, la part que le Sénat et en particulier la commission des affaires sociales ont pris dans l'examen de ces 2 réformes. Nous avons à chaque fois su prendre nos responsabilités et su faire preuve de cohérence avec nos positions passées. Qu'en sera-t-il des mesures à venir qui permettront de tenir les dépenses publiques au niveau fixé par ce programme de stabilité pourront-elles concernées de nouveau les administrations de Sécurité sociale, alors même que les besoins en matière de santé, d'autonomie sont grandissants. Ce document est assez lacunaires sur ce point essentiel, j'espère, Monsieur le Ministre, que vous pourrez nous apporter davantage de précisions à l'occasion de ce débat et je rappelle que laisser creuser la dette c'est une pure inconscience. C'est une perte de liberté. Merci. RTL. IBM. Nous entamons la suite du débat dans laquelle je souligne que la plupart des orateurs dispose d'une, d'un nombre de minutes assez restreint et qu'il serait évidemment. Préférable qu'ils s'y tiennent le 1er et monsieur Pascal Savoldelli. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Et qui est. Toujours maître de son verbe. Donc Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, l'heure est fatidique. Elle a sonné. Monsieur le Ministre, ça a été dit l'agence de notation Fitch a dégradé la note de la dette française à double aura moins, à moins. Les agences de notation vise à transcrire donc la confiance que devraient avoir les marchés financiers. Soucieux d'acquérir des obligations souveraines émises par direction générale du Trésor ou acquise sur le marché secondaire. En tant que parlementaire j'ai à m'exprimer sur la confiance. Que je place dans votre programme de stabilité que vous transmettrez à la Commission européenne. Je crois que je vous mettrai Monsieur le Ministre, d'une autre bien plus faible que double à moins. Une note plus basse, c'est comme ça et comme je constate que malgré un contexte macro-économique favorable pendant la période pré-pandémie aucune avancée majeure n'a été noté pour les services publics. Pourtant, vous l'avez répété. Et c'est même le contraire. Qu'est ce qu'on constate des déficits budgétaires importants. Et des progrès modestes sur la réduction. Et comme les agents jeudi on critique vos prévisions de croissance optimistes qui font de la perspective de réduction des déficits à 2 7 % en 2027. Les charges d'intérêts de la dette ont augmenté l'année dernière de 15 2 milliards d'euros. C'est plus que l'économie escomptée par votre réforme des retraites. Cette augmentation. Mes chers collègues, c'est un acharnement à faire plaisir aux marchés financiers et ce quoiqu'il en coûte. De fait, je cite, et là je parle de cette augmentation presque entièrement due à une augmentation temporaire des paiements d'intérêts sur les obligations indexées sur l'inflation française et européenne. Cette même indexation qui crée un qui crée en 1998 permet aux marchés financiers d'assurer leur mise. C'est quelle hérésie chercher à satisfaire à ce point les marchés financiers. Les mêmes qui aujourd'hui viennent de vous signifier leur méfiance. Vous avez décidé de faire payer l'inflation 2 fois aux Français au travers de leur consommation et en leur demandant de s'acquitter des intérêts de la dette du une nouvelle fois vous faites peser le poids de vos erreurs ont même émissaire et là on en voit la part peu parlé, mais les collectivités étant les principales mises à contribution malmenant les collectivités territoriales. C'est la société toute entière que vous malmener des territoires se retrouve, excusez-moi, mais combien de territoire se retrouve en pénurie d'eau. La désertification médicale génère colère désarroi et parfois violence, la hausse des prix, à commencer par les énergies et d'une violence faite à la dignité d'autres sujets tels que l'éducation, la sécurité, le logement, l'emploi, les transports sont également les premiers tributaire de ce que vous nous et nommer une cure d'austérité. Vous avez la politique économique hasardeuse et catastrophique, car vous ne l'emmenais pas si ce n'est au prix de déficits injustifiée et d'une dette publique qui se creuse. Est-ce vraiment aux contribuables modestes de payer les 32 milliards d'euros du bouclier tarifaire. Il y avait-il pas d'autres recettes que les seuls rente infra-marginale. Vous ne par les Français comme vous ne protégeait pas les finances publiques. Vous leur demander de payer plus tard une inflation que vous refusez de combattre. Votre gouvernement, affirme qu'un ralentissement de l'inflation alimentaire et des produits manufacturés s'observera ensuite au second trimestre. Second semestre sous l'effet des baisses passées des prix des matières premières agricoles comme industriels. Monsieur le Ministre, je suis au regret de vous rappeler une constante de l'économie qui qui peut pas vous échapper, les prix ne baissent jamais Monsieur le Ministre isolement simplement moins vite. Chaque pourcentage d'augmentation étant irrémédiable et une fois ce mensonge. Mise à jour. Alors comment pourrions-nous faire confiance. Nous n'avons eu cesse de vous alerter, en vain, de la baisse des recettes de la nation et voilà qu'un porte-parole de vos amis financiers s'inquiète à son tour de votre politique du moins d'impôts. Excusez-moi monsieur le Ministre, mais vous ne pourrez pas dire que nous, ils vont pas prévenu. Je confirme que votre réforme des retraites n'a pas rassuré. Même les marchés financiers. Et contrairement à Emmanuel Mâcon qui a invoqué dans la panique, je le cite, les risques financiers économiques trop grand pour justifier le recours à cette arme lourde anti-parlementaire 44 3 au Sénat. Les marchés financiers sont inquiets, inquiets parce qu'ils ont bien compris qu'il aura pas 17, 7 milliards d'euros d'économies d'ici 2030, mais bien moins que c'est 0 6 % de PIB pour être 8 milliards d'euros, mais inquiets surtout au regard et là je cite de l'agitation sociale qui, je vous l'affirme ne s'arrêtera pas, Monsieur le Ministre, que lorsque vous cesserez de mettre en sourdine des millions de Françaises et de Français qui se mobilisent depuis maintenant plus de 13 semaines dans notre pays. L'agence de notation estime notamment que les pressions sociales et politiques illustrée par les manifestations contre la réforme des retraites compliquons l'assainissement. Budgétaire donc plus personne vraiment ne donne crédit. Monsieur le Ministre, quand vous affirmiez pouvoir faire passer des réformes structurantes pour le père pour le pays. Plus personne ne vous donne crédit quand vous donnez des chiffres sur les effets macro-macroéconomiques de la réforme des retraites. Alors c'est vrai que les marchés financiers. Ils sont ingrats avec vous parce que vous les servez de l'autre côté il vous sanctionne, donc je vous le dis très sincèrement, il va falloir trouver un cap, pas celui de l'austérité. Il va falloir vous trouver une boussole et cette boussole ça passera pas reconnaître la légitimité sociale légitimité parlementaire merci. Très bien. La parole est ensuite à Monsieur Bernard Delcros pour l'Union centriste. Et pour quatre minutes.

Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues. Au travers de son programme de stabilité, le gouvernement affiche un objectif de réduction du déficit public ramené à 2,7% du PIB d'ici 4 ans et un ratio d'endettement public à 108,3%. Sans ambiguïté. Notre groupe partage votre objectif de réduction du déficit et de diminution de notre dette. Avec moins de 40 milliards d'euros en 2021. Plus de 50 milliards en 2022 et 70 milliards à l'horizon 2027 la facture annuelle de remboursement de notre dette s'envole et nous en connaissons les raisons. Et dans ce contexte, la poursuite de la dégradation de nos comptes publics ne peut pas être une option. Mais pour nous la trajectoire le calendrier et les solutions pour redresser nos comptes publics doivent prendre en compte plusieurs impératifs. Première réalité aujourd'hui 20% des dépenses de l'État s'engager par une loi de programmation qui prévoit une montée en puissance des crédits budgétaires de plusieurs ministères. C'est une réalité. Deuxièmement. Le redressement des comptes publics ne peut en aucun cas. Se faire au détriment des services publics essentiels dans l'État doit être garant tant de leur qualité que d'un égal accès de tous nos concitoyens. Je pense notamment à la santé, l'éducation ou encore la justice qui appelle des moyens importants. Troisièmement. Le redressement des comptes publics ne peut pas se faire au détriment des investissements qui sont absolument nécessaires pour réussir la transition écologique et technologique comme celui de la souveraineté de la France et de l'Europe dans des secteurs stratégiques. 4ème impératif la trajectoire budgétaire doit aussi intégrer les besoins des collectivités territoriales dans l'action est fondamentale pour garantir équilibres socio-économique du pays. Et ne veut pas faire non plus. Permettez-moi de l'ajouter, au détriment de l'avenir du monde rural qui nécessite la mise en Oeuvres d'une politique d'aménagement du territoire volontariste. De réussir à concilier l'objectif de redressement des comptes avec ses impératifs de dépenses et notre groupe considère que cette équation ne peut pas reposer uniquement sur la réduction de la dépense publique le levier des recettes doit aussi être. C'est d'ailleurs pour cela. Que nous avions proposé une contribution exceptionnelle de très haut, des très grandes entreprises ayant réalisé des profits exceptionnels pour financer les mesures liées à la crise. C'est aussi pour cela que nous approuvons sans réserve votre plan de lutte contre toutes les fraudes qui bien menée pourrait générer plusieurs milliards d'euros de recettes supplémentaires. De même. Je pense qu'un travail de fond en direction des niches fiscales doit être engagé rapidement. Elles représentent aujourd'hui près de 90 milliards d'euros, plus du quart des recettes de l'État et notre groupe fera des propositions dans ce sens. D'autres pistes de recettes supplémentaires pourraient d'ailleurs être envisagée. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, nous considérons qu'une coupe systématique de 5% dans les Budgets de tous les ministères de manière uniforme. Ne peut pas être la solution car elle ne permettrait pas de répondre aux besoins du pays. Ainsi, nous devons trouver un équilibre entre maîtrise de la dépense publique et c'est nécessaire. Optimisation des rentrées fiscales, il le faut et une politique de l'État au rendez vous des enjeux et des besoins du pays. Telle est pour notre groupe le défi que doivent relever les taxes. À venir et nous y apporterons notre contribution je vous remercie. Merci beaucoup. Cher collègue, la parole est à présent à monsieur Christian MILAK. Que je cherche Pardon, pardon. Il a lui-cinq minutes. Pour le groupe a simplement démocratique et social européen. Merci. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues. Je vais à mon tour participer à cette causerie. Depuis la semaine dernière, le gouvernement a rendu public le nouveau programme de stabilité pour la période 2002 3, 2027. Le Haut conseil des finances publiques a émis sa lecture des remarques. Je partage. Et ce soir le chinois va causer. Dans la sérénité et le respect. Qui caractérise notre assemblée. Que ce soit en matière d'inflation ou le taux de croissance le scénario macro et non économiques retenues par le gouvernement. Est empreint d'un optimisme hein qui n'est partagée ni par les prévisions de l'OCDE. Ni par celle de Rexecode ou devant la Commission européenne. Quant à l'Fifth elle n'est pas convaincu non plus puisqu'elle a air j'aurais réagi en abaissant la note de la France.

Je crois que la aussi. Et il y a un peu d'optimisme. Anne. Outre les ordonnances. Le gouvernement font état du retour au plein emploi en 2027 mais un tableau dans le programme de stabilité, indique que 4,5 de chômage à la même date. Je me demande quel chiffre, il faut retenir. Alors concernant ce débat je voudrais regretté que le programme de stabilité. Soit ni plus jeune ou moins que la poursuite de la politique du rabot sans réelle volonté de réformer les administrations centrales. Ces dernières continuent à doublonner dans tous les domaines avec les collectivités territoriales. Malgré la décentralisation, il y a toujours autant de ministères. Donne nos territoires les services déconcentrés de l'État sont cruellement privés de moyens. Tandis que les effectifs des administrations centrales sont soigneusement préservé. C'est ma conviction profonde. Une nouvelle phase de la décentralisation devraient être engagée au plus vite pour que l'État se consacrent pleinement à ses missions régaliennes, car à force de vouloir tout faire et les risques de tout faire mal. Je crains que les économies portent essentiellement comme cela. Était dans le fait pare-feu. La loi de programmation. Qui prévoyait un montant de 52 milliards d'euros d'efforts pour les collectivités locales. Et la sécurité sociale et peu ou prou pour l'État. Un chiffre nourri mais craignent l'excédent prévisionnel au détour d'un tableau de 0, 5. Pourcent pour les collectivités vélo cas le chiffre jamais atteint et selon moi inatteignable. Sauf sous la contrainte d'un nouveau pacte de Cahors. La prévision de l'évolution de la charge de la dette est frappante. Actuellement autour de. 40 milliards d'euros à le passerai à 49 milliards pour atteindre 75 milliards en 2027, devenant ainsi le 1er poste de dépenses de l'État. La réduction de notre dette est plus que jamais une impérieuse nécessité. En parallèle du programme de stabilité, je m'inquiète aussi. Pour 2 autres points. Nous avons connu ces derniers mois les prémices d'une crise financière mondiale. Pas de mot n'évoque ce fait radio ce scénario dans le programme de stabilité. Et j'entends aussi les annonces de l'exécutif. Avec sa volonté, vous l'avez rappelé monsieur le ministre, de baisser les prélèvements, les impôts. Je pression du CVAE. Impôts pour des classes moyennes et Entends toujours au sommet de l'État. Ne loi de programmation militaire 413 milliards. La revalorisation de chaleur de l'ingénieur. Un plan pour les urgences. Pour la justice. Pour l'industrie verte, alors où se situe les économies. En conclusion. Je dirais que ce programme de stabilité pour être fort inquiétant. Mais bien sûr. Chacun sait ici que compte qu'on a tous les programmes de stabilité, il finira au fond de l'eau tiroir bien fermée et qu'il fera vite oublier. Alors soyons rassuré. Merci, cher collègue, la parole est ensuite à Monsieur Jérôme Bascher. Pour le groupe Les Républicains. Et lui aussi pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre chargé des Comptes publics ou plutôt des comptes publics chargés. Monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues un propos liminaire et je reprendrais évidemment avec beaucoup moins de brio mais tout aussi sérieusement la remarque liminaire du président. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui commence par ne pas respecter la loi organique sur les lois de finances. Nouvellement votée. Je vous l'ai dit déjà hier en commission sur les reports de crédits. Je vous le redis ici, aujourd'hui, vous n'avez pas respecté, la dernière loi voulue par votre majorité, sur lesquels nous nous sommes accordés pour que ce pacte de stabilité soit bien transmis, 15 jours avant pour que nous puissions en discuter avant que ce soit transmis à Bruxelles, là on transmet à Bruxelles et puis après ben on vient comme dit très justement mon collègue Billac avec beaucoup de brio. À une causerie et ce n'est pas le sujet. Il s'agit bien de la trajectoire des finances publiques et donc des impôts des Français et de leur utilisation. Le rôle même et majeur du Parlement. Alors vous aviez après le toupet de dire dans ce programme de stabilité à la fin il y a un chapitre gouvernance. tous les organismes de la gouvernance sont bien là. Oubliant par là même effective en. Le. L'absence de vote sur le programme. Pluriannuel des des finances publiques. Cette loi n'a pas été voter oubliant par là même de respecter la loi organique sur les lois de finances qui elle. Le stock. Le cette bonne gouvernance. Ce n'est pas très bien. Sur la macro-économie. Le rapporteur général a été disert et a dit, oh combien effectivement vous ne prenait que les hypothèses optimistes. On n'est pas sur une trajectoire moyenne moyenne normale, on est au top surtout optimiste sur la croissance très optimiste sur l'inflation l'qu'on conseil des finances publiques le dit et le répète très optimiste aussi sur les taux d'intérêt. Tout va bien finalement. Et comme tout va bien à la fin par miracle par magie nous réussissons à passer en dessous des 3% parce que c'est la volonté actuelle de la discussion qui a lieu à Bruxelles sur la révision du parc de stabilité et des règles du pacte de stabilité. Donc on y arrive parce que on sait bien que dans la négociation actuelle hein. On n'était pas dans les clous dans la loi de programmation précédentes. C'était un peu une magie et comme la magie ne vient jamais seul. Eh bien nous avons le miracle. Pourquoi sommes-nous en dessous des 3%, c'est parce que mes chers collègues, les. Collectivités locales feront un excédent de 0 5 % du PIB qu'elles n'ont jamais fait historiquement tout à la fin, toute toute la trajectoire de croissance et l'amélioration, c'est nos finances locales qui passe de d'une amélioration de 0 1 à 0 3 puis la dernière année de 0 5 point de PIB. Autant dire que si on faisait la chose normale, c'est-à-dire autour de 0, plus 0 à moins 0 1 hé bien nous ne serons pas. Aux 3%. Nous n'y seront pas. C'est là où il y a peut être mystification et lorsque vous avez dit, le gouvernement fera un effort supplémentaire. Vous l'avez dit, vous l'avez présenté. Bah oui mais on part de pluie ou Monsieur le Ministre, on part de plus haut depuis que la dernière loi de programmation des finances publiques que nous n'avons pas voté, je le rappelle. Hé bien. Il y a 40 milliards de plus. C'est facile. De faire cela et puis effectivement ça a été souligné. Les One of. Vous les compter comment là-dedans. Comment s'est documenté parce que c'est cela qui nous a permis de passer au travers les mailles du filet à Bruxelles C'est fusil à un coup pour parler en français et One of. On les a largement utilisé. Et puis là, on ne dit plus bien comment on va faire les économies en fait ont aucune économie structurée d'ailleurs le solde structurel ne s'améliore pas. Alors il y a une bonne technique budgétaire qui consiste à expliquer dans votre programme que non bon cette année ça se dégrade encore hein. Mais alors vous allez voir, on prend de l'élan parce qu'après ça va remonter à une vitesse incroyable, non. À chaque fois qu'on dégrade, on dégrade. J'en viens enfin la dette parce que c'est quand même le coeur du du du sujet. Sur la soutenabilité. On a un énorme problème c'est on aimait aujourd'hui 135 milliards de plus. Sur les marchés à prendre, c'est énorme 135 milliards de plus parce que la Banque centrale européenne a arrêté sa politique de qui. des achats de notre dette. Donc ça il faut la passer mais le problème c'est que vous avez aussi soutenu le plan Renew You là qui. Nous envoie. 550 milliards de dettes supplémentaires. merci de la correction mais hélas ça ne corrige pas notre dette et tout ça ça fait un problème de soutenabilité parce que passer autant de dettes, il va falloir le mettre à un peu plus cher et pourquoi dans notre dette. On n'en meurt pas comme disait Oscar Wilde, mais sait-on qu'on nous on prête plus dont on meurt. Et un pays qui s'abandonne à la dette aux marchés financiers et c'est Pierre Mendès France qui le disait, c'est un pays qui s'abandonne alors moi je ne veux pas comme dirait un bon auteur qui nous manque tant que notre dette ne soient dilatée comme jamais. Très bien. La parole est ensuite à Madame Vanina Paoli-Gagin. Pour les indépendants. Et pour cinq minutes. Merci Cette annonce a fait grand bruit. Pourtant, elle ne fait que sanctionner une réalité qui ne date pas d'hier que personne n'ignore nos comptes publics sont dégradées. Ce qu'il y a de plus rageant. Avec cette décision c'est que notre pays est sanctionné pour avoir mené à bien une réforme courageuse. En mettant en lumière, je cite, l'impasse politique et les mouvements parfois violents Fitch se fait paradoxalement l'écho des opposants à la réforme. C'est avant le mal payé les efforts demandés à nos compatriotes pour contribuer au rétablissement de nos comptes publics. Le gouvernement a rappelé sa détermination totale à rétablir dans les 4 années qui viennent. Les comptes publics. Avec 2 objectifs repassé sous la barre des 3% de déficit en 2027 et réduire le taux d'endettement. Notre groupe soutient évidemment ce cap. Et c'est bien ce CAP que ce programme de stabilité dessine à grands traits. Il s'inscrit dans le prolongement des choix démocratiques qui ont été à plusieurs reprises, validé par les urnes. Il s'agit là d'arbitrage stratégiques qui doivent renouer avec une action publique s'inscrivant dans le temps long. Ce temps long, c'est celui de l'industrie, un de nos meilleurs remèdes contre la dégradation chronique de nos comptes publics. Réindustrialiser la France, c'est faire des territoires des tremplins de la relance économique dans une approche plus circulaire et plus verte et c'est accroître aussi nos employes. Réindustrialiser c'est aussi augmenter mécaniquement nos dépenses de R&D pour nous rapprocher enfin espérons-le de l'objectif de Lisbonne et trouver des solutions au problème du siècle, au 1er rang desquels la transformation écologique. Réindustrialiser cet enfin faire monter nos compatriotes en compétence pour gagner des marchés à l'export et réduire ainsi notre déficit commercial qui chaque année bat son propre record. C'est pourquoi il faut poursuivre la baisse de la fiscalité sur notre appareil productif. Continuer la suppression de la CVAE. Va dans ce sens. Il s'agit de privilégier un pilotage dynamique des dépenses et des recettes. La gestion des finances publiques est un art paradoxal souvent contre-intuitif. Baisser les impôts peut augmenter les recettes. Augmenter les dépenses pour réduire le déficit, sous réserve que ces dépenses soient effectivement génératrice de croissance à long terme. Tout est question donc de mesures et de choix stratégiques. C'est pourquoi le soutien massif et indifférencié à tous acteurs de tous secteurs n'est plus possible avec la remontée des taux le quoi qu'il en coûte n'est plus d'actualité, vous avez Monsieur le Ministre souhaiter passer oh combien ça coûte, je continue. Pour ma part de plaider pour le mieux qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte était nécessaire pour préserver notre tissu d'entreprises, soutenir les ménages pendant la pandémie. Le combien ça coûte, c'est veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Une scène exigence au vue du gonflement de notre dette provoquée par la hausse des dépenses publiques pendant la crise sanitaire. Le mieux qu'il en coûte c'est autre chose c'est optimiser le rendement de chaque euro public dépensé. Cette, cette exigence de sobriété et elle aussi impérative à moyens constants. Nous pouvons, je le pense faire mieux. Il s'agit. Puisque nous le pouvons, de le faire, nous le devons, il s'agit de redonner aux Français confiance en la puissance publique en préservant leur consentement à l'impôt. Cela passera d'abord par un audit précis et détaillé de toutes les dépenses avec des pistes de réduction vous l'avez rappelé. Monsieur le Ministre. Le gouvernement a engagé des actions pour renforcer la confiance des Français dans l'utilisation de leurs impôts. Cette confiance est indispensable pour poursuivre le travail de réformes envisagées beaucoup de chantiers restent à conduire pour éviter le décrochage productif de notre pays, alors que les géants américains et chinois sont plus que jamais et depuis quelque temps à l'offensive. Nous attendons beaucoup à cet égard du projet de loi sur l'industrie verte, nous l'avons évoqué avec notre groupe les indépendants. Cet après-midi avec les ministres le maire et Lescure l'ambition réformatrice doit rester intact pour consolider la confiance. La dégradation de la note française est postérieur à la publication du pacte de stabilité. Atteindre les objectifs proposés ne nous garantit pas du tout d'améliorer notre notre mais ne pas les atteindre risquerait à coup sûr de la dégrader encore davantage. Notre chemin et donc exigeant et ne laisse place à aucune solution de facilité. Elle ne trompe ni les Français ni les marchés. L'exemple du gouvernement trace au Royaume-Uni nous l'a récemment rappelé. Le rétablissement de finances publiques par la réduction du déficit et le désendettement et la seule voie de notre souveraineté. Monsieur le Ministre, cette voie passe pour notre groupe les indépendants par l'efficacité de la dépense publique et la réindustrialisation de nos territoires. Je vous remercie. Breuiller. Écologie solidarité et territoires et pour cinq minutes. C'est le président, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur général madame la rapporteur général, monsieur le président de la commission, chers collègues. Monsieur le Ministre vous nous transmettez avec retard, un tableau impressionniste nommé programme de stabilité 2023 2027. Moi je l'aurais intitulé baisse des déficits à l'horizon et au soleil levant. Car tout dit ton touche subtile en imprécisions choisi en lumière orienté. Vos prévisions de croissance sont estimés comme optimiste vos prévisions d'inflation sont sans doute sous-estimé et vous annoncez 5% de baisse des dépenses de l'État sans dire où ni comment vous comptez faire donc je m'interroge ou à des vous tapez sur la santé. Vous avez dit non sur le budget militaire. Non il y a une loi de programmation pareil pour celui de la sécurité. Alors sur l'éducation sur le soutien aux collectivités, il faut dire où vont se faire ces économies. Poursuivait par ailleurs une politique de désarmement fiscal de l'État par la baisse des impôts, même pour les plus aisés d'entre nous en nous privant ainsi de recettes nouvelles indispensable. Vous n'entendez pas à l'urgence écologique à sa hauteur ni la dureté de vie quotidienne des Françaises, touché par une inflation qui a atteint tout de même près de 14% entre février 2022 et 2023 selon l'Insee. Votre proposition finalement est un pack d'instabilité et un risque d'austérité. Je ne dirais pas que je suis contre la maîtrise des dépenses publiques car je sais aussi qu'il n'y a pas d'argent magique et que nous devons être vigilants sur nos dettes publiques dont le coût pèse lourd et de plus en plus lourd. Cependant, je vous le dis, la dette climatique coûtera plus cher que la dette publique. Arrêté donc les baisses d'impôts aux entreprises du CAC 40, sans contrepartie sociale ou climatiques en 2022 les bénéfices atteignent des sommets, 19 milliards pour Total énergies 11 milliards pour LVMH 23 pour CMA-CGM. 10 milliards pour BNP Paribas, les dividendes sont exponentiels, 80 milliards d'euros distribués au printemps 2022. Taxer les dividendes taxer les très hauts revenus. Monsieur le Ministre. Je crois connaître votre réponse. Nous avons déjà les prélèvements parmi les plus élevés et cette stratégie est au service de l'emploi en France hé bien je vous le dis, votre stratégie et d'abord au service des plus riches et le ruissellement n'existe pas dans la vraie vie des ménages. Trouvez-vous normal Monsieur le Ministre, que certains accumule des records de dividendes et de recettes quand d'autres peinent à se nourrir 8 sont inscrits sur la réforme des retraites d'ici 2027, c'est en gros la même somme que vous avez consacré en 2022 à la ristourne essence. Non. Limitée. Pensez-vous que ça valait vraiment le coup. Cette réforme des retraites si dur socialement n'est même pas si efficace d'un point de vue économique, tout ça pour ça. Un pays à l'arrêt pour ça. Est-ce vraiment nécessaire après la réforme de l'assurance chômage. Puis la réforme des retraites, les Français ont compris qu'au fond ce sont les droits les plus essentiels qui seront compromis pour faire des économies que le gouvernement poursuit vous allez d'ailleurs ajouté peut être du travail obligatoire pour les personnes au RSA. Tout un programme. Ces efforts se font toujours sur les mêmes créant une société où les écarts de richesse et de salaires explosent. Ça n'est pas soutenable pour qui veut une société apaisée sacraliser aussi c'est une demande le budget des collectivités territoriales afin qu'elle puisse investir et devenir les moteurs de la transition écologique et cesser de vouloir les contraindre leurs Budgets sont équilibrés. La baisse de 0 5 point exigés n'est ni plus ni moins qu'une mise sous tutelle déguisée et qui n'a pas notre agrément car les collectivités sont la clé de voûte de cette transition selon I Forcier pour être à la hauteur de la crise écologique, elle devrait vous disposez annuellement de 6 milliards et demi supplémentaire d'investissements quand quand le fonds vers les deux trains de 2 milliards d'euros sur 4 ans au risque d'ailleurs d'éparpillement d'aide mal ciblées, elles ont besoin d'investir mais ont aussi besoin d'ingénierie. C'est pourquoi nous ne comprenons pas cette volonté de rogner les ailes en contraignant le fonctionnement, laissez-les vivre le quoi qu'il en coûte, a été assumée pendant la pandémie. Il n'est plus à l'heure du jour lorsqu'il s'agit de crise climatique et pourtant, l'urgence est là et les dérèglements s'accélère. Vous savez quoi qu'en pensent les agences de notation. L'eau qui manque est plus importante que l'argent qui manque et comme dit un proverbe indien lorsqu'ils auront coupé le dernier arbre pollué la dernière goutte d'eau tué le dernier animal et pêché le dernier poisson alors ils comprendront que l'argent ne manque ne se mange pas Monsieur le Ministre. Le logiciel libéral qui contraint les dépenses publiques et par les taxations des champions du CAC 40 nous mène au chaos social et à l'impuissance climatique les 5 années qui viennent sont déterminantes pour la

qui découle d'un écart devenu abyssal entre catégories sociales et qui menacent-elles notre capacité à vivre ensemble. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame Nicole Duranton pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. dit elle dispose de 6 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues qui veut atteindre la perfection veut marcher sur l'horizon écrivait Paul Karvel dans jet d'encre en en effet l'horizon et cette ligne que nous devons garder en mire sans pour autant négliger les petits pas qui y mène. L'horizon est fixé par la trajectoire pluriannuelle présentée par le gouvernement dans le programme de stabilité 2023 2027 qui suit la ligne de l'an dernier et traduit de priorité essentielle, d'une part la nécessité de soutenir les objectifs de politique économique du gouvernement, à savoir protéger les Français face à la hausse des prix de l'énergie tout en menant des réformes d'ampleur. Il s'agit de soutenir la croissance atteindre le plein emploi accélérer la transition écologique et numérique garantir la souveraineté économique de la France et réarmer le régalien. D'autre part, la nécessité de résorber les déficits et de retrouver une trajectoire de finances publiques normalisé ce déficit public doit revenir sous le seuil de 3% à l'horizon 2027 grâce à un redressement du sol structurel de 1,3 points du PIB par an. Le poids de la dette publique commencera également à décroître à compter de 2026, ce programme détaille les objectifs qui ont été présentés à l'Automne dans la loi de programmation des finances publiques en 2022, le niveau de la dette publique s'est établi à 111 6 % du PIB, contre 112 5 en 2021 après la, l'explosion de 2020 en 2023, le ratio d'endettement continuerait sa décrue pour s'abaisser à 109 6 du PIB. Comme vous le savez, l'environnement économique international s'est dégradé à partir de fin février 2022, en raison de l'invasion russe en Ukraine, ce qui a entraîné une forte hausse des prix des matières premières, un rebond des tensions d'approvisionnement et une augmentation de l'incertitude sur les marchés en dépit de ce contexte l'évolution spontanée annuelle des dépenses publiques devrait s'établir à moins de 0,6%, l'effort annoncé cette année à 1,6% est ainsi beaucoup plus ambitieux que ceux des précédents quinquennats avec 1,4% sous Nicolas Sarkozy et un pour 100 sous François Hollande les plans tels que France relance et France 2030 permettront également de soutenir l'activité et le potentiel de croissance en préservant notre souveraineté, comme le disait notre ministre de l'économie Bruno Lemaire durant la discussion de la loi de programmation des finances publiques en novembre dernier, la France résiste mieux que ses voisins avec le taux d'inflation le plus faible de la zone euro à près de 6%. Ainsi, le gouvernement s'engage à ne pas augmenter les impôts. L'agence Fitch a certes récemment passé la note française à double à moins. Mais soyons clairs. D'une part d'autres agences comme Moody's nous a maintenus à double ah de Standard and Poor's a la France est noté plus bas que l'Allemagne et l'Autriche avec leur triple A mais plus haut que l'Espagne et le Portugal. Nous sommes dans la moyenne supérieure parmi nos voisins. Certains critiqueront en effet la dégradation de la note de la France. Néanmoins, n'oublions pas que pendant la crise Covid. Ce gouvernement a soutenu les entreprises et les ménages financière n'est pas le fruit d'une externalité subit mais bien celui d'une volonté politique bien sûr, il est possible que ces mesures ne soient pas entièrement suffisante pour soutenir une croissance économique robuste dans le contexte actuel, on peut y critiquer les limites technologiques du modèle macro-macroéconomique Mégane Pour autant les trajectoires sont fiables. Ces réformes structurelles seront également permise par de nouveaux cadres, d'une part le cadre organique français des finances publiques entrer pleinement en vigueur cette année. D'autre part le cadre européen.

on peut également noter la meilleure articulation avec les textes financiers annuels, loi de finances. Loi de financement de la Sécurité sociale et le rectificatif le Haut conseil des finances publiques peut désormais examiner la cohérence des textes financiers annuels et sectorielles au regard des objectifs de dépenses prévues en loi de programmation des finances publiques. Il faut souligner le renforcement de notre rôle en tant que parlementaire avec la présentation devant nous, d'une tragédie

la Commission européenne émet chaque année un avis sur les projets de plan budgétaire des États à l'Automne. Ces derniers sont ensuite discuté par le conseil Ecofine. Par ailleurs, ce programme sera également transmis à la commission la conformité de la France avec les recommandations du conseil sera évaluée en accord avec les dispositions du pacte de stabilité et de croissance pour faire face ensemble à ce même horizon. La Banque centrale européenne a maintenu un taux d'intérêts bas pour stimuler l'investissement de la consommation de plus l'Union européenne a mis un plan de relance de 750 milliards d'euros le groupe RDPI salue la trajectoire ambitieuse présentée par le gouvernement dans ce programme de. Stabilité et des mesures prises pour conforter le dynamisme économique en temps de crise multiple, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent monsieur Patrice Joly. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui du programme de stabilité budgétaire. Qui a déjà été adressée à la Commission européenne cette situation devient récurrente et ne peut être interprétée que comme un manque de respect de l'institution parlementaire d'autres avant moi l'ont déjà exprimé. D'un point de vue budgétaire. Il s'agit de montrer comment la France. Répond aux contraintes des règles budgétaires européennes visant à maintenir le déficit en deçà de 3% du PIB d'un point de vue politique, c'est un de. Annuel dans lequel le gouvernement. Surjoue l'orthodoxie libérale qui l'inspire auprès de la Commission européenne on arguant de sa volonté de réduction des dettes publiques. Ainsi le ministre-Lemaire martèle son souhait d'accélérer le désendettement de la France pour ramener le déficit public.

en valeur absolue. Certes, la charge de la dette, qui était de 35 milliards d'euros en 2021 et passer à 50 milliards en 2022. Vous anticipe. Et même que ce sera 70 milliards en 2027 peut être et surtout si vous poursuivez sur des réformes qui ne convainc même pas les agences de notation que vous cherchez à rassurer, voire à séduire. Avec la dette que vous brandissez, vous avez là l'argument magique pour faire peur. C'est la stratégie du choc, mise en évidence par le divorce. Peter canadienne Naomi Klein apeurés déstabilisés sidéré pour avancer sur ses objectifs. Or si vous préciser que cela représente 1,5% du PIB ou de 3% des dépenses publiques en 2021 nov du PIB en 2022 de 2% du PIB en 2027, cela fait à juste titre beaucoup moins peur. Faut-il rappeler que la hausse de 15 milliards de charges de la dette en 2022 a été principalement le fait des missions croissant de titres de dette indexée sur l'inflation. Que rien ne justifie économiquement mais qui bien sûr protège les revenus financiers des détenteurs de la dette d'État comme parallèlement vous répéter toujours la même antienne baisser les recettes fiscales et les cotisations sociales au nom de la compétitivité. Tout cela ne peut conduire qu'à une réduction drastique des dépenses publiques tout particulièrement des dépenses sociales et des services publics. Vous envisagez ainsi de réduire les dépenses publiques de 0 8 % en moyenne en volume par an. Donc 0 5 pour les collectivités locales, or ici. Tous les ans on a ici tous les ingrédients d'une austérité qui va enfoncer notre pays dans l'impasse. Rendons au passage les objectifs économiques, sociaux et écologiques inatteignable. Il est utile de noter que l'affront que disait déjà l'an dernier. Quelle chance 2030 il faudra mettre sur la table 22. Entre 22 et 100 milliards d'euros. Pour assurer la transition environnementale. Encore faudrait-il rappeler que le point important de la dépense lui. Français s'explique d'abord par son modèle social et fiscal qui prend en charge les dépenses essentielles en matière de santé de retrait d'éducation que d'autres pays relever du secteur privé ensuite d'une démographie plus dynamique en enfin d'un budget de la défense. Conséquent dont vous avez annoncé l'augmentation. Alors Monsieur le Ministre, au nom de la réduction de la dépense publique doit-on abonné de notre système français de protection sociale et de services publics auxquels les Français sont très attachés parce il croustille tu le Patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nos services publics sont-ils en si bon état. Qu'il faille réduire les moyens qui leur sont alloués, êtes-vous sourd à la détresse des territoires la détresse sanitaire de nombreux territoires, doit-on se plaindre d'avoir une démocratie plus dynamique. Souhaitez-vous revenir sur le budget défense réduire massivement le poids de la dépense publique ne peut se faire sans modifier la qualité de vie des ménages et la capacité à agir des collectivités locales. Il y a de quoi s'inquiéter à fortiori lorsqu'on sait

Le nouveau monde promis en 2017. Ne constituerait-t-il part en fait à appliquer les vieilles recettes. Thatchérienne et nous faire revenir 40 ans en arrière, alors même qu'investir dans les transitions est de nature à renforcer la stabilité la solidité financière de la France en. Enfin, Monsieur le Ministre si le FC autre obsession est vraiment la dette. Dans ce cas, augmenter les impôts des plus riches et supprimer de nombreux allégements fiscaux dont le montant global s'élève depuis 2017 et dans la perspective des quatre années qui viennent, à 364 milliards, c'est-à-dire plus qu'un budget annuel du du pays comment encore cautionner que les 370 ménages aux revenus les plus élevés, est un taux effectif d'impôt sur le revenu de l'ordre de. 5% avoisinants. Même les 0,26% pour les 37 familles les plus riches, selon l'économiste Gabriel Zucman dont l'expertise vient de plus être. Par la prestigieuse médaille de John Bates Clark pour conclure et sans surprise, ce sont encore les classes moyennes et populaires. Ils continueront à faire les frais du libéralisme économique que vous mettez en place depuis 2017 avec les risques démocratique que l'on peut percevoir. Je vous remercie. Très bien. La parole est à présent à monsieur Vincent Capo Canellas autres questeurs pour l'Union centriste et pour quatre minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame et monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues. D'abord une remarque de méthode. La question je crois n'est pas de faire le procès du gouvernement ou de telle ou telle la question et que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus les mains, les moyens de tergiverser, car nous n'avons plus les marges de manoeuvre. Vous avez compris monsieur mais ce qu'il fallait très vite recalée le discours et la pratique. Vous avez commencé à est le discours, il nous faut et, il vous faut recaler la pratique. Pour autant, la question de savoir si ce que fait le gouvernement et. Celle-ci elle est pleinement légitime. Elle est même salutaire car cette fois, nous avons la pression des taux et des marchés. Non pas tant que les marchés des des laisse notre dette mais parce qu'il tests que les annonces qui sont faites maintenant. Ne soit pas éventuellement vérifier demain et il y a là-dessus quelques points dollars. Ce débat sur le programme de stabilité, l'occasion de rappeler l'attachement de l'autre groupe à la maîtrise des comptes publics ce cap sur lequel le gouvernement se projette aurait sans doute pu, il aurait dû être plus volontariste, la volonté de rétablissement des finances publiques qui annoncé dans ce programme. En revanche, nous regrettons le manque de précision quant au modus operandi. La dépense publique n'est pas mauvais en soi. Lorsqu'elle est utilisée à bon escient et les crises récentes l'ont montré. L'argent magique n'existe pas et les fonds employés devront être remboursés. La condition de notre souveraineté. Tient en 2 mots le sérieux budgétaire. Force est de constater que dans la ville et du au comité des finances publiques, cela a été rappelé à un certain nombre de points d'alarme existe des prévisions de croissance pour 2023. Optimiste, ça a été dit. Des prévisions de croissance effective. Relevé. Reposant sur une hausse de la consommation des ménages nettement supérieure à celle enregistrée avant la crise du Covid. Tout cela pose quand même quelques questions. Vous avez décidé de fonder vos, vos prévisions sur des hypothèses avantageuses, cela a été déjà rappelé notamment une croissance potentielle de 1 35 % jusqu'en 2027, alors même que le scénario de la Commission européenne envisagée dans le cadre de la réforme de la gouvernance européenne évidence public qui est beaucoup moins favorable. L'incertitude autour de votre scénario demeure donc élevé, dans un contexte international plus voulons que jamais où les incertitudes sont encore nombreuses. L'évolution des cours internationaux des matières premières et l'énergie, le niveau des taux d'intérêt et la fragilité des marchés financiers constituent les aléas majeur. Cela a été dit par notre collègue Bernard Delcros, la volonté de contenir les dépenses de doit pas aussi con conduire à des coups de rabot uniforme que ce qui serait à la fois injuste, inefficace. La France va se doter d'une vraie stratégie d'évaluation de hiérarchisation des dépenses à laquelle le Parlement. Cela a été rappelé notamment par le président de la commission et le rapporteur général doit être pleinement associés. D'un côté vous assurer tout mettre en oeuvre pour maîtriser le budget de l'autre les crédits des ministères augmente. De 24 milliards et la charge de la dette tutoie les 60 milliards en 2023. Une fois neutralisé la baisse des dépenses exceptionnelles engagées en réponse aux crises. La dépense publique hé bien prévu en hausse en volume il y a un point qu'il faudra regarder de plus près l'objectif annoncé dans ce programme de stabilité ne saurait substituer à une. À une loi de programmation qui fait actuellement défaut. Cette loi de programmation des finances publiques doit être adopté au plus tôt et ça sera rassurant pour tout le monde. Elle devrait afficher une trajectoire crédible de réduction de la dette publique reposant sur des hypothèses macroéconomiques réalistes et une stratégie claire et documentée de maîtrise de la dépense publique, il n'en reste pas moins bien sûr que les points de satisfaction existe au milieu du groupe Union centriste. Le gouvernement enfin pris la mesure de l'urgence pour la France de se désendetter en révisant ses objectifs à l'horizon 2027, la signature de notre pays sur les marchés doit demeurer crédible cette crédibilité n'est pas indéfectible l'abaissement par l'agence Fitch d'un cran de la note de la France est un 1er signal d'alerte afin de préserver notre crédibilité. Nous devons intensifier nos efforts et vite. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le rapporteur général a très bien exprimé l'optimisme du gouvernement sur le calcul des divers indicateurs à rebours des analyses extérieures. L'abaissement de la note de la France par l'agence Fitch vient nous pousser à mener un peu plus une véritable politique d'assainissement des comptes publics. Désormais, outre les Français nous allons devoir convaincre le reste de la planète que nous pouvons accéder à la trajectoire proposer. Notre groupe rapport rappelle depuis des années dans cet hémicycle. La nécessité pour l'État de s'engager dans une démarche sincères de rétablissement des comptes publics. Ce processus doit devenir impérativement réalité. Nous vous avions alerté sur des risques à fonder votre politique sur la dette avec les nouveaux taux la charge de notre dette ne cessera. De croître pour quasiment doubler d'ici 2027. Nous sommes par conséquent très sceptique sur le réalisme de la trajectoire envisagée. Le recours à une prévision de croissance et un des flatteurs jugée unanimement excessif nous portes à craindre que vous soyez obligé d'agir sur des variables d'ajustement. Aussi je voudrais ici évoquer dans ce contexte particulier le traitement des collectivités locales, d'autant plus qu'elles auront à entrer dans le processus de la transition énergétique. Vous prévoyez en effet que leur soldes s'améliorera la faveur de la poursuite des efforts de maîtrise de la dépense de fonctionnement et vous tablez en matière d'investissements sur une baisse en fin de période grâce au cycle électoral la trajectoire proposé elle là aussi optimiste. Dans votre analyse, vous comptez sur l'inflation pour réguler les hausses en volume, sachant que par ailleurs la plupart des recettes sont désormais aux mains de l'État depuis le passage à une fiscalité d'impôts nationaux. Vous escomptez donc un effet des taux en un seul mot Inflation Fiscalité réguler pour compléter le dispositif. Vous envisagez une association des APUL à l'effort de modération de la dépense publique en concertation avec les divers avec Exit l'article 23 de la programmation précédentes. Et les contrats de Cahors avec un effort de ralentissement moindre de 0,5% demandés aux collectivités par rapport au, 0 8 % de l'État. Dont acte. Mais nous nous interrogeons à cet égard sur les mécanismes de la concertation auquel il sera recouru. Cas ainsi que nous l'avons maintes fois évoqué dans cet hémicycle. Les conditions d'une concertation ne sont pas réunies. Le passage à une fiscalité nationale entièrement ordonnancer par le gouvernement et la persistance d'une fiscalité locale comme d'un système de financement obsolète. Laisse totalement entre les mains de l'État la conduite la négociation. Qui peut procéder. À sa guise À sa guise au coup par coup. Or, sans vouloir un retour chimérique car l'autonomie fiscale. Il nous semble primordial qu'un nouveau processus permet aux collectivités de retrouver une libre-administration cela ne passera que par une réforme réelle de la fiscalité et des dotations sur des brasses cohérente et contemporaine en tenant compte à la fois des charges des et des besoins des territoires comme des dynamiques locales. Cette réforme est urgente l'exigera pour vivre une double articulation au plan national entre l'État, les autres sous secteur et au niveau interne entre les collectivités elles-mêmes aussi elle doit introduire une nouvelle gouvernance du système qui sera l'espace de dialogue et de concertation attendu réunissant l'État le Parlement les collectivités. C'est seulement à ce prix que nous réintroduire on la libre administration propre à une démocratie moderne. Faute de cela le programme de stabilité demeurera pour nous à un pacte léonin. Pour nous faire changer d'avis, il conviendrait que nous disposions après échéance d'une loi de programmation intégrant au moins l'ébauche d'un tel dispositif. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre attention. À cet égard. Merci, cher collègue, la parole. À présent, madame Monique Lubin. Le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances. Le programme de stabilité, qui fait l'objet du débat qui se tient aujourd'hui confirme que le gouvernement persiste à creuser son sillon néo-libérale. Il s'est inscrit en effet dans la droite ligne du projet de loi de programmation des finances publiques et que le Parlement a refusé d'adopter en novembre 2022. Le président du Haut Conseil des finances publiques n'a d'ailleurs pas manqué de s'émouvoir dès janvier 2023, du fait que la France demeure dépourvue de ce texte crucial prévu par la Constitution. Comment en effet concevoir des politiques publiques sont que soit anticiper un plafond global des dépenses de l'État sur le périmètre de la norme de dépenses et des plafonds de dépenses par mission. Saisie par le gouvernement du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale portant réforme des retraites. Le Haut Conseil a d'ailleurs relevé que l'absence d'adoption du projet de loi de programmation des finances publiques ne lui permettait pas de vérifier la cohérence des prévisions de finances publiques des textes financiers avec la loi de programmation. Cette loi de programmation rejetée par les assemblées s'inscrivaient elles-mêmes et comme il se doit dans la droite ligne du programme de stabilité soumis par l'exécutif en avril 2022 aux institutions européennes qui ne tiennent qui ne tiennent pas, rappelons-le, le stylo du gouvernement. Or que trouver ton dans le programme de stabilité d'avril 2022, un projet de réforme des retraites avancées par l'exécutif français pour répondre à des objectifs macro-économique selon son scénario, le recul de l'âge de départ à la retraite doit d'abord accroître le taux d'emploi des Français en favorisant l'emploi des seniors. Il n'est pas question de sauver le système des retraites. Nous avons amplement démontré lors des débats sur la loi de finances rectificative, l'absurdité de la démarche. Qui des portera les dépenses vers d'autres branches de la Sécurité sociale. Ce qui conduira à l'échec à venir du gouvernement concernant le 2ème objet objectif affiché la réduction du déficit de l'État. Cet objectif n'est pas poursuivi sérieusement, comme en témoignent les baisses d'impôts consenties aux plus riches et aux grandes entreprises. Sur la dernière décennie, l'exécutif a ainsi organisé la perte annoncée de 372 milliards d'euros de recettes, soit une moyenne annuelle de 37 milliards par an. Ces chiffres sont à rapprocher de l'hypothétique déficit du système de retraite de 13 milliards et demi d'euros pour 2030 que le gouvernement prétend chercher à prévenir dans le même temps les économies espérées du report de l'âge légal de la retraite à 64 ans sont de 8 milliards d'euros en 2027 soit le strict montant du cadeau fiscal qu'est la suppression de la CVAE. Pour mémoire, le Fonds monétaire international a lui-même signalé en octobre 2022, à la France que ces baisses d'impôts ne sont pas opportune, mais le gouvernement s'en-tête. Ce qui est cohérent avec une ligne politique identifiable depuis longtemps et notamment avec la stratégie retenue pour gérer la dette Covid n'a-t-il pas fait endosser cette dernière à la protection sociale par le biais de la cadet alors que le quoi qu'il en coûte n'a pas été une politique sociale mais bien une politique économique. À Sciences Po Paris. Le mois dernier d'éminents spécialistes ont déploré que la réforme des retraites s'inscrivent dans le cadre d'une politique macro-économique il y a été redit qu'une réforme des retraites reflète un projet de société et ne peut être une variable d'ajustement pour la réduction des déficits. Ne nous y trompons pas. Arbitrage il y a eu de la part du gouvernement qui a tranché pour sacrifier 2 ans de la vie des Français les plus vulnérables et en faveur de la baisse de la dépense publique plutôt que de la préservation et de l'accroissement de la ressource. Les collectivités sont d'ailleurs également concernés par ce refroidissement annoncer de la dépense publique et la menace d'un retour de la contractualisation. Mais c'est un autre sujet. Ces choix le gouvernement les paie aujourd'hui dans la rue. Mais les Français les paient encore davantage et de bien des manières par une crise démocratique dangereuse pour la nation par une crise sociale par la dégradation même de la note de la France pour l'emprunt sur les marchés financiers. Monsieur le Ministre quand tirerez-vous les conclusions de la crise dans laquelle nous a plongé. Votre gouvernement. Sous le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous avez présenté le 27 avril dernier, la nouvelle ligne budgétaire de la France jusqu'à 2027 et nous allons ce soir en quelque sorte commenter une orientation déjà transmises. Pour réduire la dette, vous comptez vous appuyer notamment sur des économies de dépenses sans vraiment les documenté et alors que le quoi qu'il en coûte persiste ainsi la crédibilité du dispositif reste donc interrogé avant que la revue des dépenses soit engagée et le cap et que le cap soit clair. Est-ce que cela allait rassurer les agences de notation qui réexamine le cas français et la Commission européenne qui promet un retour à des règles budgétaires plus contraignantes. L'an prochain, même si elles pourront être différencié. Visiblement non. Fitch qui a été le premier à se prononcer vient de dégrader la note de la France. Notre situation budgétaire et ses déficits miroir 160 milliards d'euros budgétaire et autant commercial inquiète tous les Européens. La réforme des retraites était un 1er gage économie au mieux entre 7 et 10 milliards déjà démenti par ex aequo d'. Cet exercice en constitue un ce. Un second. Mais tout cela est-il vraiment crédible. Ce n'est pas vraiment gagner, on le voit déjà les nouveaux objectifs budgétaires plus ambitieux pour le quinquennat, sont indispensables mais doivent être réel une nouvelle trajectoire qui promet un désendettement plus rapide et bien sûr nécessaire mais manque cruellement de concret. En dévoilant les grandes lignes du programme de stabilité, le document envoyé tous les ans à Bruxelles et gravant dans le marbre les prévisions budgétaires sur 5 ans. Malgré l'absence d'une loi de programmation de nos finances publiques. Que vous nous annoncez maintenant pour cet été. Vous reconnaissez enfin la situation de bascule, celui de la fin de l'argent gratuit. Reprendre le contrôle de notre dette pour garder le contrôle de nos choix et enfin de poser le cadre indépassable de l'action publique. Il était temps. Dans le détail vous promettez maintenant de ramener le déficit à 2 7 % du PIB en 2027 alors qu'il était encore des. Cette fin 2022 et qu'il est prévu, désormais à 4, 9 fin 2023. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport aux précédentes prévisions qui tablaient sur 2, 9 en 2027. Ce que nous réclamions dès 2022 au niveau de la commission des finances du Sénat est enfin retenue. C'est surtout sur la dette. Que vous voulez le plus offensif. Celle-ci doit être ramené à 108,3% du PIB en 2027, affirmé vous c'est vraiment un minimum. À l'Automne. L'objectif était fixé à 119, c'est mieux. Et pourtant encore bien timide et surtout insoutenable. J'ai trouvé d'ailleurs un peu osées que vous fassiez des comparaisons européennes alors que notre niveau et 1,8 fois supérieur à celui de l'Allemagne. Les taux d'emprunt remonte à grande vitesse depuis quelques mois et promettent d'alourdir le coût de la dette que notre notation revue à la baisse va encore accélérer nous le dénonçons depuis au moins 2 ans. La charge de la dette devrait atteindre plus de 71 milliards d'euros en 2027 et représenté à cet horizon le 1er poste de dépenses de l'État. Ce constat est posée depuis longtemps et le déni ne peut plus durer. Notre politique budgétaire ne peut pas passer par des hausses d'impôts qui viendrait casser la faible croissance. Voilà un point d'accord. D'un, au contraire, il s'agira ensuite et seulement ensuite après avoir baissé la dépense d'amorcer une baisse de nos prélèvements obligatoires car non seulement notre dépense publique est exorbitante. Mais en plus elle est inefficace. Il suffit de voir la situation de nos services publics en milieu rural, par exemple pour comprendre la grogne et l'incompréhension. Où va notre argent. Voilà la formule lapidaire, la plus répandue dans les échanges que nous avons avec nos concitoyens. Récemment, la Cour des comptes, comme d'autres, avait évoqué un scénario économique optimiste pour qualifier vos hypothèses de croissance potentielle d'ici à 2027. Le Haut conseil et sur cette même ligne dans son avis, bien évidemment. Quant à l'effort d'économies il serait demandé à l'État une baisse de ses dépenses de 0 8 % en moyenne par an hors inflation et ce dès l'an prochain mais où et comment. Point d'interrogation. Quid de la réduction de la dépense fiscale. Point d'interrogation. Surtout ne nous répondez pas que ce sera sur le dos des collectivités territoriales. Elles ont déjà beaucoup donné et ne sont en rien responsables de la situation budgétaire de notre pays au contraire elles un assurent l'essentiel de l'investissement pendant que l'État emprunte toujours plus pour fonctionner. Et pourtant, il semble bien que ce soit grâce à elle que vous franchissez l'obstacle des 3% en 2027. Vous l'aurez compris ce programme ne nous convient pas. Nous craignons même que vous ne continuez à jouer avec des allumettes. Alors que nous sommes assis sur un volcan. Je vous remercie. Et après ce dernier orateur des groupes. La parole est à nouveau au ministre délégué. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénatrices et les sénateurs je veux d'abord. Commencer par remercier chacune et chacun des intervenants pour leurs interventions le remercier par ailleurs d'être resté pour écouter. Ma réponse aussi tardivement dans la soirée. Je vais essayer de répondre à chacune et à chacun en tout cas sur les points principaux sans pour autant faire traîner nos débats à des heures indécentes. 1er point d'abord sur le calendrier, ça été abordées notamment par les sénateurs Bachere est joli non. Ce programme de stabilité n'a évidemment pas été transmis à la Commission européenne avant d'être présenté au Parlement. Et c'est au moins le mérite de ce débat que de le clarifier, nous respectons la. Procédure le programme de stabilité et transmis à la Commission européenne. À l'expiration du délai de 15 jours après sa transmission au Parlement. Il sera donc transmis à la Commission européenne postérieurement à ce débat. Il y aura donc un tout léger retard avec les délais demandés par la Commission européenne, puisque nous devons théoriquement transmettre le programme de stabilité avant le 30 avril. On aura donc quelques jours de retard à mettre en perspective avec les quelques mois de retard que nous avions eu l'an dernier, du fait de la séquence électorale de la présidentielle et des législatives. Je crois que c'était près de 3 mois et demi de retard là ce sera une dizaine de jours beaucoup de mieux mais en tout cas on respecte, évidemment la procédure, il n'est pas question de transmettre ce programme de stabilité à la commission avant que le Parlement se sent soit. Saisi, je précise par ailleurs que nous avons fait le choix du fait de l'examen de la réforme des retraites d'attendre que la réforme des retraites soit définitivement adopté et validée par le Conseil constitutionnel et promulguée pour que le programme de stabilité soit présenté. Je pense que sinon nous on aurait pu nous le reprocher d'anticiper sur l'adoption de cette réforme majeure évidemment pour notre trajectoire avant de la présenter toujours sur les questions. De calendrier, je confirme, comme l'a dit la Première ministre, que la loi de programmation des finances publiques sera représenté à l'été un petit point de correction cependant parce que j'ai entendu dans certaines interventions que ce texte aurait été rejeté par les assemblées. Non, le Sénat a adopté une loi de programmation des finances publiques qui n'est certes pas celle qui avait été présenté par le gouvernement, mais il y a eu un texte adopté au Sénat et la discussion va se poursuivre sur cette base. Le 2ème, point sur lequel je veux revenir qui est ressorti des débats.

Je ne dirais pas que notre macro-économie. Et optimiste ou que nos prévisions de croissance par exemple sont optimistes. Je dirais qu'elles sont volontaristes. Volontariste. Et je crois que nous avons eu raison d'être volontariste dans nos précédentes prévisions. Moi je me souviens quand même à l'été dernier, quand on prévoyait une croissance de 2,5% pour l'année 2022, on nous a dit vous êtes démesurément optimistes bah on a eu raison d'être volontariste puisque la croissance en 2022 a été de 2,6 de la même manière à l'Automne dernier quand un certain nombre de prévisions prévisionniste prévoyez une récession dans la zone euro une croissance atone, voire nul. En France, on nous a accusés d'être optimiste avec une prévision de croissance à 1% pour l'année 2023 nous avons assumé d'être volontariste. Et je pense que nous avons eu raison de le faire parce que depuis le mois de janvier, les prévisionnistes revoient tous à la hausse leurs prévisions qui se rapprochent les unes après les autres de la prévision de croissance à 1% du gouvernement pour l'année 2023. Le FMI est à 07 aujourd'hui. L'OFCE à zéro huit ces prévisions sont beaucoup plus proches des nôtres, que celle qui avait été fait à l'Automne dernier là aussi nous avons eu raison d'être volontariste sur la croissance. Potentielle dans ces travaux de l'Automne, le Haut conseil des finances publiques tablait sur une croissance potentielle entre 0 9 et 1 3, du fait de l'incertitude de certaines réformes avec un 35 par an. Nous sommes proches, très proches de la fourchette haute du HCFP présenté à l'Automne dernier. Je rappelle que l'évaluation de la croissance potentielle est aussi proche de celle du FMI, qui est à 1 3 est proche de celle de la Commission européenne au moins sur le court terme 2022 2023 qui est à un 4. Je veux rappeler ensuite qu'un certain nombre de prévisionnistes n'ont pas tenu compte de l'ensemble des réformes qui figure dans notre programme pour évaluer la croissance. Potentiel sur les années à venir et d'ailleurs une partie des prévisions qui avaient pu être faites ces derniers mois ne tenait pas encore ton compte de l'impact de la réforme des retraites, encore moins de la réforme à venir du RSA évidemment dans nos sous-jacent sur nos prévisions de croissance potentielle. Il y a le programme de réformes, sur lequel nous nous sommes engagés qui vise à atteint de la société du plein emploi. Jusqu'à présent nous avons montré que nous tenions les engagements que nous avons pris de ce point de vue là, nous avons fait la réforme de l'assurance chômage. Nous avons fait la réforme des retraites, nous ferons la réforme du RSA. La réforme du lycée professionnel qui aussi auront un impact sur l'activité dans notre pays sur l'emploi, sur l'activité économique et donc sur la croissance potentielle, un point rapide. Ce qu'on pourrait en parler assez longtemps. Sur le déflecteur du PIB qui a été mis en avant, notamment par le rapporteur général. En 2022. Le déflecteur du PIB avait été nettement moins dynamique que prévu. Nettement moins dynamiques que les prix à la consommation du fait du choc des termes de l'échange liées au conflit en Ukraine qui a entraîné côté demandent des prix d'importation nettement plus dynamique que les prix d'exportation et donc une contribution fortement négative des prix du commerce extérieur côté offre un prix de valeur ajoutée comprimés par le délai de transmission de la hausse des prix d'entrants au prix de vente en 2023 effectivement le des flatteur et révisé à la hausse pour résorber cet écart. Il s'établit ensuite de manière cohérente avec l'inflation au sens de l'IPC. Donc, là où le précédent stable tablait sur une convergence lente du déflecteur du PIB et de l'inflation au fil du quinquennat. Il est désormais fait l'hypothèse et c'est cohérent au regard des dernières observations macro-économique d'une convergence rapide sur 2023 2024, toujours sur ces questions de conditions macro- économique, une réponse à la question de la rapporteure générale Doineau qui m'a demandé quel impact pouvait être mesurée de la dégradation par l'agence Fitch sur nos conditions d'emprunt, comme l'a dit à Bruno Lemaire tout à l'heure aux questions au gouvernement. On peut qualifier cet impact de limiter à ce stade, puisque nous, nous avions un écart avec l'Allemagne un spread comme on dit, de 57 points de base vendredi, juste avant l'annonce de Fitch. Cet après-midi Bruno Lemaire a dit nous sommes passés à 59 donc c'est plus de et, ce soir nous sommes même à 58. Donc plus hein donc c'est un impact qui est. Mineur et je réponds aux sénateurs Sautarel qui a indiqué que l'agence Fitch était la première à réévaluer la notation souveraine de la France. Non puisqu'il y a eu l'agence Moody's, la semaine dernière qui n'a pas réévaluer la notation de notre pays en là maintenant donc à la notation précédentes je viens ensuite sur. Un autre point qui est celui des choix politiques et budgétaires qui sous-tendent ce programme de stabilité, le premier choix effectivement que nous faisons, c'est celui de l'emploi et du travail et je remercie les sénatrices Paoli-Gagin et Duranton d'avoir insisté sur ce point là ça passe effectivement par la baisse de certaines fiscalité oui nous l'avons assumé. Nous avons assumé sur un certain nombre de points dans le précédent quinquennat de vouloir ramener notre pays. Proche de la moyenne européenne. S'agissant de la pression fiscale sur les entreprises et sur l'activité économique pour libérer l'emploi s'il n'y avait pas eu d'impact en matière d'emploi. Je pourrais entendre et même comprendre des critiques fortes sur ce choix là. Mais la réalité c'est que nous avons créé plus d'1.500.000 emplois en Net dans notre pays que le taux de chômage au plus bas depuis 15 ans le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans, c'est donc bien qu'il y a eu un impact sur ce sujet et je réponds aux sénateurs jolie qui a à parler des allégements de cotisations sociales. Les allégements de cotisations sociales sont aussi favorables à la création d'emplois mais d'ailleurs la gauche le sait puisque je rappelle que sous le gouvernement de Lionel Jospin et la gauche plurielle. Les allégements généraux de cotisations ont doublé et ça a eu un impact sur la création d'emplois dans notre pays qu'on vous fait baisser le coût du travail. Mécaniquement vous libérer la possibilité d'embaucher et d'employer pour nos entreprises, qu'il s'agisse des plus grandes ou des PME. TPE donc effectivement nous avons fait ce choix et nous l'assumons. Nous avons fait ce choix et nous avons alors c'est un débat qu'on a régulièrement des recettes supplémentaires, alors même que nous avons baissé certains tôt on collecte plus d'impôt sur les sociétés depuis que le taux est à 25% qu'à l'époque où le taux était à 33% ensuite. Des baisses d'impôts qui ciblent les ménages ou les particuliers. J'ai entendu un certain nombre d'interventions, notamment monsieur. Brouillé et Madame Lubin. Si on parlait de baisse d'impôts pour les plus riches, les très riches. vous avez pas parlé de nantis mais bon voilà les des plus riches. Très sincèrement, moi je suis absolument persuadé que dans votre département du Val-de-Marne, que ce soit à cinq morts à Alfortville à Fontenais ailleurs quand vous croisez des Français qui sont désormais exonérés de taxe d'habitation ou de redevance télé. Je ne crois pas qu'ils vous disent que ce sont des nantis ou des très riches. Pourtant ce sont eux qui ont bénéficié de la grande majorité des baisses d'impôts pour les particuliers que nous avons consentis, c'est cette classe moyenne qui travaille et qui a toujours le sentiment que quand il y a des dépenses publiques de notre modèle social ou quand il y a des baisses de fiscalité, ça ne lui bénéficie jamais. Et moi je crois qu'avec ces mesures, elle a trouvé à voir qu'elle pouvait aussi être soutenu si vous conjuguer les deux, en moyenne, taxe d'habitation et redevance télé c'est autour de 1000 euros sur l'année pour tous ces Français. Je n'imagine pas qu'on vous les croisez que vous parlez de ces baisses d'impôts, vous les qualifiez de nantis ou de très riches, pourtant c'est la très grande majorité des baisses d'impôts, en volume, ce sont pour ces Français. Qui travaille ces français de la classe moyenne que nous voulons soutenir. Ensuite le deuxième choix que nous faisons, après celui de l'emploi et du travail, c'est celui de l'investissement dans nos services publics et là je vraiment répondre à Monsieur Savoldelli. On ne peut pas dire qu'il y a une forme de désertion budgétaire des services publics. Quand le budget de l'hôpital public dépasse les 100 milliards d'euros. Quand on prévoit cette année. 4 milliards 700 millions d'euros de plus pour l'éducation nationale. Moi je me souviens en 2012 quand François Hollande est élu, il annonce un grand plan de réinvestissement pour l'éducation nationale, un milliard 500 millions d'euros de plus sur l'année 2013, on fait 4 milliards 700 millions d'euros de plus sur l'année 2023 avec des revalorisations salariales inédite depuis le début des années 90 pour nos enseignants sur la défense. Le budget de la Défense dans notre pays 2017 versus 2027, c'est plus 75% il y a jamais eu un tel effort de réinvestissement sur un temps si court pour notre défense dans notre pays sur la question de la justice depuis 2017, le budget a augmenté de 42% sur la police pour citer d'autres exemples, nous faisons des choix de réinvestissement dans nos services publics, mais comme l'a dit monsieur Sautarel. Et je le rejoins totalement. L'enjeu c'est pas seulement combien on dépense, c'est comment on dépense, c'est pas seulement de dépenser plus, c'est de dépenser mieux. Et là c'est l'enjeu majeur des réformes qui sont portées doivent être portées par mes collègues et il en va de même pour la transition écologique et moi je veux répondre aux sénateurs que pour moi il n'y a pas à choisir entre les 3% et les 3 degrés. Que si on veut régler la question de la transition écologique, ça nécessite des investissements. Et si on veut pouvoir investir, il faut avoir des conditions de financement qui nous permettent de le faire et si on veut avoir des conditions de financement qui nous permettent de le faire, il faut être responsable et sérieux avec la dépense publique pour être capable d'emprunter, de faire les bons emprunt qui sont vertueux pour la transition écologique et qui nous permettent d'investir et qui permettent aux collectivités. Local de le faire, elles sont absolument essentiels pour cela. Je viens d'ailleurs au sujet des collectivités locales

parce que ça n'a pas lieu, se trouvait dans le pays stable ce sera dans la loi de programmation des finances publiques en tout cas en proposera de le mettre dans la loi de programmation des finances publiques, avec effectivement la traduction et ça a été soulevée par le sénateur. Que désormais, nous demandons un effort de maîtrise des dépenses plus important à l'État qu'aux collectivités locales, 08 pour l'État en volume versus 0 5 pour les collectivités locales en volume là où dans la précédente copie les collectivités locales, il aurait été demander un effort supplémentaire mais qui dit et fort ne veut pas dire saigner. Moi je veux quand même insister sur le fait qu'avec cette trajectoire. Les collectivités locales dépenseront en 2027 pour leur fonctionnement. Plus de 13 milliards de plus que ce qu'elles dépensent aujourd'hui, on est loin de l'austérité, loin de la saignée dans les dépenses publiques, on parle simplement de se fixer collectivement. Une règle consistant à dire qu'on cherche à maîtriser la progression de nos dépenses de fonctionnement. Et sur la question de savoir comment on va le faire, qui a été posée, notamment par le sénateur gainé. On y travaille avec les associations d'élus dans le cadre de la des assises des finances publiques, on en est à la 2ème ou 3ème réunion au niveau technique entre nos services et les associations d'élus, on les a par ailleurs reçu avec Bruno Lemaire. Moi j'ai bon espoir que nous trouvions un moyen de nous accorder. Sur la manière dont nous pourrons maîtriser la progression de nos dépenses publiques. L'autre moyen de. D'atteindre notre trajectoire. C'est également aussi de lutter contre la fraude et je veux vraiment remercier le sénateur Delcros d'avoir insisté sur ce point là c'est vrai que l'an dernier nous avons eu une année. 14 6 milliards d'euros de droits notifiés suite aux contrôles fiscaux de la direction générale des finances publiques. 800 millions d'euros de redressement. Sur le volet social par les Urssaf. C'est une année historique pour le saluer faut saluer tous les agents qui concourt à ces résultats. Et évidemment, l'objectif du plan fraude que je présenterai dans les prochains jours auquel vous avez très largement contribué puisque tous les groupes de cet hémicycle étaient représentés. En tout cas est invitée à être représentés dans le groupe de travail que j'ai mis en place ont pu porter des propositions et je pense se retrouveront dans une bonne partie d'entre elles, l'objectif c'est effectivement aussi d'améliorer nos recettes par ce biais là et je serai très attentif, vous l'avez dit monsieur Delcros aux propositions de votre groupe pourra faire sur la question des niches fiscales, c'est un enjeu sur lequel je crois on a tous la volonté d'avancer, c'est quand on rentre dans le détail que ça devient plus difficile. Mais cela nécessite qu'on y travaille ensemble. effectivement, c'est une trajectoire ambitieuse. Ça a été dit par le sénateur Sautarel et je veux vraiment le remercier. J'ai entendu quand même dans beaucoup d'interventions la reconnaissance que ce programme de stabilité est nettement plus ambitieux que celui que nous avions présenté l'an dernier qui était en sous-jacent à la loi de programmation des finances publiques de l'année dernière 4 points de dette en en moins en 2027 que dans la précédente copie un déficit lui aussi revu à la baisse en 2027 par rapport à la précédente copie l'enjeu c'est d'y arriver ensemble et je pense que nous pourrons y arriver ensemble. Moi je souhaite qu'on puisse continuer à travailler. Il en, il y a eu l'an dernier une initiative. Était nouvelle, elle était pas parfaite. On a un peu essuie les plâtres mais je pense qu'elle a eu certains mérite en tout cas ça a été reconnue par un certain nombre de parlementaires y compris des oppositions c'est les dialogues de Bercy et je souhaite réitérer cet exercice des dialogues de Bercy cette année en version améliorée et enrichie en commençant plus tôt avec davantage d'échanges et davantage de données qui pourront être communiquées par mon ministère à l'ensemble des parlementaires qui en font la demande, on prie pour chiffrer certaines propositions que vous pourrez faire ou certaines économies que vous seriez amenés à proposer, je pense et nous l'avons vu dans les interventions que les enjeux sont majeurs pour notre pays. Il justifie, je crois que nous avancions tous ensemble de concert pour ma part, j'y suis prêt. Merci à tous. Je vais lever la séance. Prochaine séance jeudi 4 mai à 10h 30 pour le débat sur le thème comment rendre possible le retour en Ukraine des enfants déportés en Fédération de Russie. La séance est levée.